La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 24 octobre 2019 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation

Cette école républicaine, qui trouve son socle dans les lois Ferry de 1881 et 1882, a pour objectif de former des citoyens à la République et de les intégrer dans la société. C'est la raison pour laquelle je fais miens les propos de Jules Ferry, dans sa lettre de 1883 aux instituteurs et institutrices sur l'école laïque, tendant à établir la neutralité confessionnelle des écoles : Sans doute [le législateur] a eu pour premier objet de séparer l'école de l'église, d'assurer la liberté de conscience et des maîtres et des élèves, de distinguer enfin deux domaines trop longtemps confondus, celui des croyances qui sont personnelles, libres et variables, et celui des connaissances qui sont communes et indispensables à tous, de l'aveu de tous. » Plus tard, dans sa circulaire du 15 mai 1937, Jean Zay, ministre de l'éducation nationale, soulignait à son tour l'importance de la neutralité de l'école républicaine, en précisant : « Ma circulaire du 31 décembre 1936 a attiré l'attention de l'administration et des chefs d'établissement sur la nécessité de maintenir l'enseignement public de tous les degrés à l'abri des propagandes politiques. Il va de soi que les mêmes prescriptions s'appliquent aux propagandes confessionnelles. L'enseignement public est laïque. Aucune forme de prosélytisme ne saurait être admise dans les établissements. Je vous demande d'y veiller avec une fermeté sans défaillance. quinze ans, la loi interdisant le port de signes religieux ostentatoires dans les écoles publiques françaises, voulue par le président Chirac, était adoptée par le Parlement.

Il était devenu indispensable de permettre à nos enfants d'acquérir des savoirs dans l'harmonie garantie par la République française, afin de préserver leur liberté de conscience. Depuis lors, la question de la neutralité des accompagnants des sorties scolaires refait régulièrement surface,

mis fin à cette polémique : « Il est recommandé de rappeler dans le règlement intérieur que les principes de laïcité de l'enseignement et de neutralité du service public sont pleinement applicables au sein des établissements scolaires publics. Ces principes permettent notamment d'empêcher que les parents d'élèves ou tout autre intervenant manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions religieuses, politiques ou philosophiques lorsqu'ils accompagnent les élèves lors des sorties et voyages scolaires. Ainsi était affirmée la nécessité de l'absolue neutralité des parents concourant au service public de l'éducation en participant aux sorties scolaires et astreints, de ce fait, au respect des valeurs fondamentales du service public français, au premier rang desquelles le principe de laïcité. Un principe, du reste, partagé à droite comme à gauche, si bien que Vincent Peillon décida de ne pas abroger la circulaire Chatel, après l'élection de François Hollande à la présidence de la République. Plus tard, sitôt nommée, Najat Vallaud-Belkacem déclarait que l'acceptation de la présence d'accompagnatrices voilées lors des sorties scolaires devait être la règle et son refus, l'exception. Cette position peu claire a conduit les juridictions à adopter des positions contradictoires à travers la France, laissant aujourd'hui les enseignants face à un vide juridique insécurisant, sans principe unique régissant les sorties scolaires. En juillet dernier, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé que le principe de laïcité imposait que les personnes participant à des activités assimilables à celles des personnels enseignants à l'intérieur des locaux scolaires soient astreintes aux mêmes exigences de neutralité. Par ailleurs, il apparaît clairement à toute personne douée d'un minimum de bon sens que les sorties scolaires font partie intégrante du temps scolaire et s'inscrivent dans le cadre du service public de l'éducation.

Il est primordial de veiller au respect de la liberté de conscience des élèves, principe fondamental reconnu par les lois de la République, affirmé par l'article 1 de la loi du 9 décembre 1905, et de tout faire pour éviter qu'ils ne soient, du fait de leur vulnérabilité, des proies pour tous les prosélytismes. Comme le faisait observer Lionel Jospin, alors ministre de l'éducation nationale, dans une circulaire de 1989, « rien n'est plus vulnérable qu'une conscience d'enfant ». Et de préciser Les scrupules à l'égard de la conscience des élèves doivent amplifier, s'agissant des enseignants, les exigences ordinaires de la neutralité du service public et du devoir de réserve de ses agents. Il convient de rappeler que les sorties scolaires constituent des temps d'activités pédagogiques destinés aux élèves et non à leurs parents, qui n'ont en aucun cas l'obligation d'y participer. De fait, l'accompagnement des sorties scolaires est proposé aux parents, sur la base du bénévolat ; il doit, dès lors, s'inscrire dans le respect des principes régissant le service public de l'éducation. Tout parent désireux d'accompagner une classe dans le cadre d'une sortie doit donc se soumettre au principe de neutralité déjà imposé par la loi aux enseignants et aux enfants. Devant le vide juridique auquel nous nous trouvons confrontés, mais surtout face aux graves menaces pesant sur notre unité et le respect d'un des principes qui la fondent, la laïcité, le législateur ne peut pas rester passif.

Cette disposition de bon sens, largement adoptée par le Sénat, n'a malheureusement pas été retenue par la commission mixte paritaire. Par ailleurs, la Fédération des délégués départementaux de l'éducation nationale elle-même, à l'occasion de son congrès de juin dernier, a adopté une motion demandant la reconnaissance de la fonction d'auxiliaire bénévole du service public de l'éducation pour les personnes accompagnant les sorties scolaires, ce qui entraînerait pour ces personnes une obligation de neutralité et de respect de la liberté de conscience des enfants. des enfants. Voilà pourquoi j'ai déposé, le 9 juillet dernier, en dehors du contexte médiatique actuel et de toute polémique, une proposition de loi, cosignée par un certain nombre de nos collègues, tendant à assurer la neutralité religieuse des personnes concourant au service public de l'éducation.

Les collaborateurs occasionnels du service public étant, pour l'heure, considérés comme de simples usagers de celui-ci, l'adoption de cette proposition de loi permettra d'étendre à ces personnes l'exigence de neutralité religieuse dans l'exercice de leur mission bénévole auprès des élèves.

Il nous revient aujourd'hui, dans cet hémicycle, de défendre l'héritage de Jules Ferry et de Jean Zay, en affirmant haut et fort notre détermination à protéger l'innocence et la liberté de conscience des enfants dans un pays secoué par des tensions politico-religieuses. Il s'agit non pas d'un combat entre la droite et et la gauche, mais d'un combat républicain, rien d'autre. Car, comme l'a souligné Robert Badinter, la laïcité est « une grande barrière contre le poison du fanatisme Tous les enfants que nous accueillons dans nos écoles sont des enfants de la République, qui doivent pouvoir vivre et s'épanouir en dehors de toute tentative d'influence, sans être les otages de pressions politiques ou religieuses. Nous avons à former les citoyens de demain dans une école où ils doivent être accueillis avec sérénité et apaisement, sur un socle commun : la République une et indivisible

dans le contexte politique et médiatique qui préside à l'examen de la proposition de loi de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio, il me paraît important, pour que nos débats gagnent en sérénité, qu'ils se concentrent sur l'école, et elle seule,

à l'ancien professeur d'histoire que je suis de revenir brièvement, pour peser et pour poser les choses, sur ce qui caractérise, depuis l'origine, notre école publique. Pour ses pères fondateurs, l'école avait une mission essentielle : permettre à l'élève de se construire librement en tant que citoyen, à l'abri de toute influence extérieure. Cet idéal émancipateur a eu immédiatement un corollaire : la neutralité de l'école publique face aux croyances. Ainsi, dès 1882, le cours d'instruction religieuse devint leçon d'instruction morale et civique.

les signes religieux furent progressivement retirés des salles de classe. Ce contexte historique fondateur rappelé, mon cours d'histoire achevé ... Quittons donc le XIX siècle pour en venir à la situation actuelle, en posant quatre questions nécessaires à un débat serein. Première question : qu'est-ce qu'une sortie scolaire ? Les circulaires de 1999 et 2011 sont claires. Celle de 1999 précise : « Les activités pratiquées à l'occasion d'une sortie scolaire viennent nécessairement en appui des programmes. Elles s'intègrent au projet d'école et au projet pédagogique de la classe. Chaque sortie, quelle qu'en soit la durée, nourrit un projet d'apprentissages. » J'en veux pour preuve l'interdiction faite aux élèves, depuis la loi de 2004, de porter des tenues et signes religieux ostensibles non seulement dans le bâtiment scolaire, mais aussi lors des sorties scolaires. L'application de cette loi par le ministre de l'éducation nationale le montre : les sorties scolaires sont bel et bien du temps scolaire. Elles doivent donc être neutres du point de vue des croyances religieuses. Deuxième interrogation : que signifie, justement, la neutralité du point de vue des croyances à l'école publique ? En la matière, le législateur s'est progressivement montré particulièrement strict. Ainsi le droit impose-t-il une neutralité religieuse dans l'enseignement public aux personnels, comme dans tous les services publics, mais également aux usagers que sont les élèves, mineurs ou majeurs, depuis la loi de 2004, qui a restreint leur possibilité d'afficher leurs croyances religieuses- une loi simple, peu bavarde et finalement parfaitement acceptée et appliquée.

depuis la décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 juillet dernier. Mes chers collègues, le service public de l'éducation est donc l'unique service public qui impose à ses usagers- en l'occurrence, les élèves -une restriction de la manifestation de leurs croyances religieuses. En somme, les intervenants à l'extérieur des salles de classe, donc les accompagnants de sorties scolaires, sont désormais les seuls à ne pas être soumis, dans les activités liées à l'enseignement, à ce principe de neutralité religieuse ou,, à une à une restriction de la manifestation ostensible de leur appartenance religieuse. Or qu'est-ce qu'un accompagnateur ? C'est là ma troisième question.

Participant à une activité scolaire, le parent devient un accompagnateur [ ...] Il contribue ainsi à la bonne marche de l'activité pédagogique. Il a donc un devoir d'exemplarité devant tous les élèves concernés par cette activité, dans son comportement, ses attitudes et ses propos. » Mes chers collègues, j'insiste : dans son comportement, ses attitudes et ses propos. Ajoutons qu'il paraît important de traiter cette question aussi du point de vue de l'enfant. En effet, il me semble difficile de croire qu'un enfant de 4 ans, ou même de 8, serait capable de faire la subtile différence statutaire et réglementaire entre l'accompagnant et l'intervenant. Pour lui, il s'agit dans tous les cas d'un adulte, qu'il doit écouter et vers lequel il peut se tourner en cas de problème. à l'heure de la coéducation et de l'inclusion des parents dans la communauté éducative, à l'heure où les fédérations de parents d'élèves souhaitent que ceux-ci deviennent davantage encore des partenaires à part entière de l'école, considérer le parent d'élève une sortie scolaire comme un simple tiers me paraît paradoxal. Sauf à penser que le parent serait un acteur en tout, sauf pendant la sortie scolaire, où il devrait rester motus et bouche cousue ! Non, il s'agit bien d'un collaborateur occasionnel du service public, bénéficiant d'ailleurs de ce statut en cas d'accident pendant l'activité. Pour autant, une loi est-elle nécessaire ? Telle est ma quatrième question. Je le crois sincèrement, afin de clarifier une situation qui n'est pas acceptable pour les directeurs d'école et les chefs d'établissement.

Le Conseil d'État indique que le parent d'élève est un simple usager du service public de l'éducation, non soumis, donc, au principe de neutralité religieuse il demande à l'autorité compétente de déterminer si « des considérations précises relatives à l'ordre public, au bon fonctionnement du service public d'éducation ou à la nature des missions confiées aux parents » justifient l'application du principe de neutralité à l'adulte accompagnant la sortie scolaire. C'est là que naît l'inconfort juridique, qui rend une loi Au reste, plusieurs syndicats de chefs d'établissement et d'inspecteurs, lors de leur audition, nous ont fait remarquer que, en l'absence de textes clairs, les directeurs apprécient seuls les considérations mentionnées par le Conseil d'État,

l'article 1 de la loi de 1905, une loi de liberté, affirme que la République protège la liberté de croire ou de ne pas croire

: c'est s'en prendre à ce que des hommes considèrent comme sacré ; par là, c'est s'en prendre à la République, protectrice de la liberté de conscience. Nous examinons cet après-midi la proposition de loi

Je pensais d'ailleurs que nous en resterions là ... Je regrette d'avoir à revenir cet après-midi sur ces sujets. Pour moi, la situation est claire. Lorsque j'ai dit, récemment encore : « pas interdit, mais pas souhaitable », je n'ai fait que résumer la situation actuelle.

C'est le trésor de notre République que de nous donner, avec la laïcité, les clés de la liberté en même temps que de la concorde nationale. C'est une question qui appelle discernement et esprit de responsabilité.

concerne une activité non située dans l'espace scolaire, mais qui relève du temps scolaire ; il concerne l'encadrement des élèves par des adultes, mais qui ne sont pas des fonctionnaires. Selon l'angle choisi, on peut défendre l'un ou l'autre des points de vue. Le respect du principe de laïcité s'impose à l'ensemble des personnels du service public. À ce titre, il leur est interdit de manifester des convictions religieuses, notamment par le port de signes religieux ostentatoires.

doit-on les considérer comme des usagers ou des collaborateurs occasionnels du service public ? Le Conseil d'État, dans son étude de 2013, a rappelé que la manifestation des convictions religieuses avait pour limite le trouble à l'ordre public ou au bon fonctionnement du service public.

s'agissant des parents d'élèves qui participent à des déplacements ou des activités scolaires, à recommander de s'abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses

entraîne un risque de prosélytisme ou de pression inacceptable sur les élèves. Bien sûr ! Une loi qui interviendrait en la matière irait au-delà du nécessaire et aurait des effets contre-productifs. Elle irait au-delà du nécessaire, parce qu'elle poserait en règle absolue ce qui relève du discernement quotidien. Il est impossible de demander à la loi de réglementer chaque aspect de la vie courante

En allant au-delà du nécessaire, une loi serait aussi contre-productive, parce qu'elle enverrait un message brouillé aux familles. C'est ce qu'on disait en 2004 ... Nous voulons rapprocher les familles des écoles : c'est la meilleure chance d'accomplir le projet républicain.

nous devons envoyer aux enfants le message que les parents sont les bienvenus, et que c'est ensemble, parents et école, que nous assurons leur éducation. C'est ainsi que nous pouvons compter sur une contagion positive des valeurs de la République. L'école, c'est l'espace de la science, de l'argumentation, du discernement. L'enfant a besoin d'un cadre de neutralité pour forger ses convictions et son esprit critique, ... Précisément ! ... dans la plus belle tradition philosophique et scientifique de notre pays. L'histoire de l'école républicaine témoigne de cette volonté collective de mettre nos enfants à l'abri des passions des adultes.

qui reste une référence pour nous tous. Il écrivait que l'école doit « rester l'asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas ». La laïcité, avant d'être un principe qui s'impose à tous, fut à la racine de l'école de la République.

En 1882, un enseignement laïque est institué dans les écoles primaires. La morale religieuse est remplacée par l'instruction morale et civique. Nous sommes vingt-trois ans avant les lois de 1905. Nous aurions eu peut-être à l'époque des débats inversés entre les travées qui se trouvent à ma gauche et à ma droite ... En 1886, la loi Goblet confie à un personnel exclusivement laïque l'enseignement dans les écoles publiques. La loi de 2004 interdisant le port de signes ostentatoires à l'école s'inscrit dans cette longue tradition républicaine. C'est une loi de clarté qui fait aujourd'hui largement consensus. On le voit bien : cette laïcité est notre héritage commun. Elle devrait être ce qui nous unit totalement sur l'ensemble de ces travées. Comment mieux le rappeler qu'avec les statues qui m'environnent ? Ce n'est pas seulement 1905, ce n'est pas seulement 1881, ce n'est même pas seulement 1789 qui ont préparé la laïcité. C'est le long travail des siècles qui a permis de faire la distinction entre ce qui relève du divin, et donc de la conscience de chacun, et ce qui relève du politique, c'est-à-dire des règles communes à tous. C'est Michel de L'Hospital, qui nous met en garde contre les risques de la discorde. C'est Malesherbes, qui s'est battu pour la liberté de pensée dans un esprit d'équilibre, en nous gardant de tout excès. C'est Molé, qui a su se lever contre des lois injustes.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je n'ai jamais pensé que la laïcité était un principe du passé. Je crois au contraire qu'elle est un principe profondément moderne. Ce que nous voulons avec la laïcité, c'est l'application concrète de l'idéal républicain. Cet idéal républicain est un idéal d'émancipation de chacun par l'éducation,

et qui ne correspond pas à ce que nous entendons par République : des sociétés qui préfèrent juxtaposer des communautés plutôt que de faire vivre le contrat social entre des citoyens égaux. Ces sociétés dont nous ne voulons pas courent le risque de la fragmentation. Très bien ! Ce sont des sociétés qui souvent aujourd'hui s'interrogent sur leur devenir. Ils sont nombreux, nos cousins, en Europe ou même ailleurs,

La laïcité est un trésor français. Elle se traduit par un corps de règles. Ce corps de règles, j'ai tenu à le préciser dès mon arrivée au ministère de l'éducation nationale. Ce n'est pas un ministre inactif en matière de laïcité qui est devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs. Si ! Nous avons établi un vade-mecum de la laïcité qui est à la disposition de l'ensemble de la communauté éducative. Il établit à partir de cas concrets ce qu'il convient de faire. Nous avons mis en place des équipes laïcité mobilisées dans chaque rectorat pour intervenir au cas par cas dans chaque établissement, chaque fois qu'un personnel de l'éducation estime qu'on a contrevenu au principe de laïcité. Du vent ! Par-delà tous les discours, ce sont des centaines d'interventions qui ont eu lieu depuis deux ans dans les établissements

Jour après jour, je me tiens personnellement informé des écoles et des établissements dans lesquels le contenu des enseignements ou le comportement du personnel va au-delà de ce qui est acceptable. Avec la loi pour une école de la confiance, vous avez aussi voté il y a quelques mois le contrôle de l'instruction à domicile, qui est désormais renforcé. De surcroît, par l'article même loi, vous avez permis l'interdiction de tout prosélytisme aux abords des établissements scolaires. Merci ! C'est un apport considérable qui aura des effets très importants dans les temps à venir. Voilà des mesures concrètes. Nous n'avons pas besoin de grands débats pour nous épuiser. Nous avons besoin, concrètement, d'assurer un équilibre entre des positions et, surtout, de lutter contre le communautarisme, contre la radicalisation et pour la laïcité.

Parce qu'elle est indivisible, nous combattons fermement toutes les tentations de repli communautaire. Parce qu'elle est laïque, nous veillons à éduquer nos enfants dans un espace de raison, hors de toute emprise, quelle qu'en soit la nature. Parce qu'elle est démocratique, nous luttons sans relâche contre toutes les idéologies qui prônent l'inégalité. Enfin, parce qu'elle est sociale, nous offrons le meilleur à chaque enfant, quelle que soit son origine, et nous portons une attention constante aux plus fragiles pour les amener au plus loin de leur talent. Voilà la République que nous souhaitons au XXI siècle. Voilà le cap que nous devons toujours garder pour notre école. Redonnons du sens au mot « laïcité », redonnons du sens à notre destin collectif. Ce dernier a un nom : la République ; il a un objet l'émancipation de tous ; et il a une raison d'être qui nous unit : notre pays, la France

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je voudrais tout d'abord vous dire, monsieur le ministre, que vous avez très bien parlé. Maintenant, il faut passer aux actes

73 % des Français souhaitent l'interdiction du voile islamique ou des signes communautaristes ostensibles pour les parents qui accompagnent les sorties scolaires-c'est l'objet de la présente proposition de loi et 72 % des Français souhaitent que l'employeur puisse interdire les signes religieux ostensibles pour les salariés du secteur privé. Ce sondage confirme, d'une part, que cette proposition de loi est la bienvenue et qu'elle répond à un besoin et à une aspiration de nos concitoyens,

Ce constat m'amène à déposer la présente motion de renvoi à la commission. En effet, la commission aurait pu manifestement compléter de manière utile et constructive le texte initial. initial. Il faut dire clairement non à tout ce qui peut favoriser de près ou de loin le terrorisme islamique. Il faut donc dire non à la radicalisation et non à toutes les formes de communautarisme islamique. Il faut aussi dire non à certains flux migratoires, au sein desquels le terrorisme essaie de recruter. À ce sujet, je pose une question pourquoi les migrants de religion islamique viennent-ils se réfugier en Europe et pas dans les pays musulmans, pourtant voisins, d'autant que certains de ces pays sont particulièrement riches et ont les moyens financiers de les accueillir ? De même, pour quelle raison les bateaux prétendument humanitaires accueillent-ils les migrants immédiatement en limite des eaux territoriales de la Libye

sont juridiquement sûrs au sens du droit international et qu'ils sont beaucoup plus proches que les ports français. Par le passé, les immigrés qui venaient en France voulaient s'intégrer dans nos sociétés. Aujourd'hui, les flux migratoires sont différents ; ils conduisent à la formation de noyaux communautaristes qui rejettent notre façon de vivre. Les personnes immigrées ou issues de l'immigration ne doivent pas nous imposer leurs us et coutumes. Au contraire, si les intéressés viennent dans notre pays, c'est à eux de s'adapter à notre mode de vie et aux règles de notre société.

et félicité l'élu de la région Bourgogne-Franche-Comté qui avait protesté lors d'une séance du conseil régional contre la présence, dans le public, d'une femme voilée accompagnant la sortie scolaire de jeunes enfants.

les jeunes enfants, car il est très dangereux pour un jeune enfant d'être confronté tout petit à des actes et à tendances communautaristes radicalisantes. C'est dans cette logique que j'ai déposé trois groupes d'amendements sur le texte que nous examinons. Le premier vise à interdire le port du burkini et l'organisation d'horaires séparés pour les femmes dans les piscines.

si vous êtes musulman ou de telle ou telle religion, vous avez le droit de faire ce que vous voulez : vous pouvez les laisser agoniser dix minutes dans un coin, il n'y a pas de problème ! Quel est le rapport ? Il y a des

la France réglemente l'abattage des animaux de boucherie, qui doivent être étourdis avant d'être tués. Malheureusement, il y a ces dérogations qui entraînent de longues agonies des animaux.

le contraire de ce que vous venez de faire à la tribune en important tous les débats de la société, toutes les querelles des hommes dans l'école, parce que, comme je le disais en conclusion de mon intervention, la conscience des enfants,

la proposition de loi sur la neutralité religieuse lors des sorties scolaires est inscrite au débat de notre Haute Assemblée. Avant même d'être discutée, elle a déjà fait l'objet de nombreux débats dans les médias ou dans l'opinion publique. Permettez-moi, pour commencer, d'essayer de l'analyser au-delà de toute polémique et en faisant abstraction dans un premier temps du contexte dans lequel elle intervient. L'encadrement législatif et réglementaire actuel est-il suffisant, ou y a-t-il un trou dans la raquette juridique ou une imprécision qui nécessiteraient un nouveau dispositif législatif ? Telle est la question qui nous est posée par cette proposition de loi. Pour notre part, nous l'abordons avec le souci de préserver l'esprit de la loi de 1905 et également de celle de 2004, qui-doit-on le rappeler ?-sont des lois d'équilibre dont le fondement ne doit pas être remis en cause. De ce point de vue, il est utile de rappeler que le voile, comme toute autre tenue inspirée par la religion, à condition qu'elle ne trouble pas l'ordre public, n'est pas interdit en France. Son usage, en revanche, est encadré, notamment pour préserver la neutralité dans les services publics et protéger l'enfant dans l'école alors que sa conscience n'est pas encore formée.

Indéniablement, ce dispositif nous paraît perfectible. La proposition de loi apporte de ce point de vue deux améliorations notables. la décision d'accepter ou pas des parents en fonction de leur tenue lors des sorties scolaires relèvera non plus du directeur d'école, mais de la loi. À bien des égards, d'autant plus compte tenu des débats actuels, il semble en effet préférable de ne pas faire reposer cette décision sur les seuls directeurs d'école. Dans certaines villes, nous pouvons du reste nous interroger pour savoir s'ils ont réellement le choix, actuellement, d'accepter ou de refuser tel ou tel parent. Deuxièmement, les sorties scolaires participent clairement de l'activité pédagogique et, à ce titre, la notion d'école hors l'école introduite par un amendement du rapporteur précise de manière utile leur situation juridique. permet d'interdire que l'élève arbore un signe ou une tenue ostentatoire lorsqu'il sort de l'école pour participer à une sortie scolaire. Dans l'état actuel du droit, rien ne s'y oppose. la proposition de loi ne nous semble pas apporter une clarification suffisante sur le statut d'accompagnant. Ce dernier n'a en effet jamais été défini, si ce n'est en creux, à travers des jurisprudences. Un statut permettrait clairement de préciser la mission qui incombe à l'accompagnant et sa responsabilité. Il s'agirait ainsi d'établir la différence entre l'enseignant ou l'animateur, qui, à travers la pédagogie utilisée, participe clairement d'une activité d'enseignement, et l'accompagnant, dont la mission est uniquement de permettre que la sortie ait lieu. S'agissant du risque de prosélytisme et de la nécessité de protéger l'enfant, il nous semble que mettre sur le même plan l'intervenant et l'accompagnant est inexact. L'un participe de manière active et directe à l'enseignement, l'autre n'a pas, en revanche, vocation à y prendre part. De ce point de vue, la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Lyon, qui porte sur l'intervenant, ne peut être complètement utilisée pour justifier la proposition de loi actuelle. Nous sommes également en droit de nous interroger pour savoir si le caractère bénévole permet d'assimiler les parents accompagnateurs à des collaborateurs occasionnels du service public ou à des usagers. Le Conseil d'État, en 2013, a répondu à cette question de manière claire en leur attribuant le statut d'usagers. Je ne peux m'empêcher de rappeler que, du point de vue du risque de prosélytisme qui doit nous préoccuper, les sorties scolaires ne méritent sans doute pas d'être devenues en quelques semaines le symbole d'une intrusion dangereuse de la religion dans l'école. Nous devrions être plus inquiets des phénomènes plus pernicieux et dangereux pour les jeunes que sont le développement de l'instruction à domicile et celui des écoles hors contrat, dès lors qu'ils ont pour objectif de soustraire complètement les enfants à l'enseignement de matières comme les sciences ou l'histoire par les écoles de la République pour les placer sous le joug d'un obscurantisme religieux. Nous le voyons à travers cette rapide analyse : la proposition de loi apporte des réponses utiles, mais qui ne sont que partielles tant que le statut de l'accompagnant n'est pas clarifié. Mais l'essentiel n'est peut-être pas là. Nous ne pouvons en effet faire abstraction du contexte dans lequel ce débat intervient. L'emballement médiatique de ces derniers jours a mis sur le même plan la question du port du voile lors des sorties scolaires, la présence de listes communautaires aux élections municipales et même, comme cela a été évoqué récemment, l'interdiction de signes ou de tenues ostentatoires dans l'espace public. Dans ce grand déballement commencé par un élu écervelé du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, un peu de raison et de sérénité s'impose. Notre assemblée gagnerait à ne pas se laisser happer par ce tourbillon en se saisissant à tout prix de ces sujets, en multipliant les propositions de loi ou en créant des commissions d'enquête. Disons-le franchement, pour un certain nombre d'entre nous, ce qui gêne dans cette proposition de loi n'est pas tant le contenu que le contexte dans lequel celle-ci intervient, un contexte où les amalgames simplificateurs prennent le pas sur les discours raisonnés, où la voix des modérés est peu audible par rapport à celle des extrêmes et où les réserves des uns ont peu de poids face à la récupération politique des autres. Ce contexte appelle à la prudence et à la réserve. La crainte est forte en effet que cette proposition de loi ne fasse qu'alimenter le débat tel que nous le connaissons depuis quelques jours, sans y apporter la sérénité nécessaire. Est-ce la vocation du Sénat d'y participer dans ces conditions ? Absolument ! Sur les sujets sensibles face auxquels l'angoisse du temps présent fait l'objet d'une exploitation par des extrémismes de tout poil, nous gagnerions collectivement à prendre plus de recul et à témoigner pour rappeler simplement ce qu'est notre histoire et ce qui fonde notre concorde nationale. Dire cela, c'est faire preuve non pas d'angélisme ou de laxisme, mais de lucidité pour identifier ce qui pose problème et ce qui n'en pose pas.

et de ses lieux de culte, en suggérant d'améliorer la formation par la création d'un conseil scientifique unique chargé de la définition d'un programme commun, ou en proposant un meilleur financement du culte musulman. C'est encore ce que le groupe Union Centriste a fait en faisant voter la proposition de loi de notre collègue Françoise Gatel pour mieux encadrer les écoles privées hors contrat. Le sujet n'en était pas moins délicat, bien au contraire ! Mes chers collègues, nous le savons, la voie est étroite entre la nécessité de lutter avec force contre le communautarisme et la radicalisation,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a de grandes lois auxquelles il ne faudrait jamais toucher, tout du moins en ce qui concerne les valeurs qu'elles portent, comme la loi de 1905 dont les articles 1 et 2 posent les fondements de la laïcité. Selon ces articles, en effet, « la République assure la liberté de conscience » et « ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Malheureusement, il y a aussi des lois opportunistes, mal faites et mal pensées, que l'on est contraint d'examiner : c'est le cas du présent texte. Vous prétendez vouloir sortir du flou qui entourerait l'accompagnement des sorties scolaires par les mères voilées et combler ainsi un vide juridique qui serait devenu manifeste. C'est faux Aujourd'hui, la jurisprudence administrative est claire et limpide : les parents accompagnateurs sont des usagers du service public de l'éducation et, en tant que tels, ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité qui incombe aux agents publics et qui dépasse, d'ailleurs, la seule sphère religieuse. Seulement, ce postulat, pourtant d'une logique implacable, ne vous convient pas. Vous essayez donc de tripatouiller la loi, afin qu'elle entre en résonance avec votre idéologie- pardonnez-moi l'expression, mais je n'en trouve pas d'autres quand je vois le texte de la commission

lors que l'on commence à lui accoler des épithètes, c'est que l'on s'éloigne de son sens originel et qu'on la vide de sa substance pour mieux y substituer sa propre conception. Exactement ! Mes chers collègues, la laïcité n'est pas une palette chromatique dans laquelle chacun choisirait sa coloration en fonction de sa sensibilité. La République a magnifiquement défini la seule et unique laïcité qui existe, c'est-à-dire la possibilité laissée à chacune et à chacun de croire ou de ne pas croire dans un esprit de concorde et de tolérance mutuelle. Robert Badinter l'a récemment présentée comme l'« une des grandes barrières contre le poison du fanatisme, parce que vous reconnaissez l'autre tel qu'il est, comme tel qu'il est, comme humain, avec les mêmes droits que vous, quelle que soit sa religion. [ ...] C'est l'autre que je rencontre dans le respect ». Évidemment, la laïcité interroge avant tout notre rapport individuel et collectif à l'altérité, la manière dont nous parvenons ou non à vivre en société. Elle est cette pierre angulaire sur laquelle repose notre socle commun. Et il est terrible de constater que c'est en son nom, que c'est en l'instrumentalisant que d'aucuns effritent progressivement ce socle et finissent par fragmenter et déliter la communauté nationale ! Immigration, islam, communautarisme, radicalisation, tout est amalgamé, parfois sciemment. Et ce désordre alimenté en permanence empêche de régler les vrais problèmes et dérives qui se font jour, puisque tout n'est que confusion. Arrêtons de tout mélanger et de tout confondre ! Oui, la République a sûrement des territoires à reconquérir, mais il s'agit d'un sujet d'une nature et d'une ampleur tellement différentes et tellement plus importantes que celui qui nous occupe actuellement. Interdire aux mères voilées d'accompagner des enfants lors de sorties scolaires pourrait se révéler contre-productif et ne fera qu'ériger un fossé entre la République et ses citoyens de confession musulmane. La laïcité exige une éthique de responsabilité. Or, dans le cadre de ce texte, je ne l'aperçois pas. À l'opposé des fondamentalistes qui prospèrent sur le sentiment d'exclusion, et à l'opposé des identitaires qui ne peuvent accepter une société multiple, nous ne voterons pas cette proposition de loi. sagesse, mes chers collègues, le Sénat ayant pour tradition de prendre de la hauteur et de viser l'apaisement, surtout dans le contexte actuel. Ne nous trompons pas de combat en faveur de la laïcité, ne nous trompons pas de combat en faveur de la République, ne la desservons pas ! Comme s'exclamait Aristide Briand, nous n'avons pas le droit de faire une loi qui ébranle la République. Très Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, une actualité récente donne à l'examen du texte de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio un écho particulier, dont nous nous serions bien passés. Cette proposition de loi s'inscrit en fait dans le prolongement de la discussion du projet loi pour une école de la confiance,

dans lesquelles certains se sont depuis engouffrés. Tirant les conséquences de cet épilogue, notre collègue a déposé sa proposition loi en juillet dernier. Nous ne pouvions alors imaginer que deux événements médiatiques déclencheraient la frénésie. Il y tout d'abord eu la polémique récente autour de l'affiche de la FCPE. Elle a pris à contre-pied nombre d'observateurs qui connaissent bien cette fédération, dont les statuts sont pourtant depuis toujours de nature laïque. La seconde polémique fait suite à la provocation absurde d'un élu du Rassemblement national, qui ne connaît apparemment ni les règles d'accueil du public dans l'enceinte de sa collectivité ni le droit de cette mère d'élève à accompagner une sortie scolaire en l'état actuel des textes. Cette forme d'humiliation envers une maman devant son enfant est humainement inacceptable ! Si la question de l'expression religieuse des accompagnants de sorties scolaires n'est pas nouvelle, aucune solution concrète n'a jamais été trouvée ni dans la loi ni dans les circulaires Royal ou Chatel encore en vigueur. On le voit bien aujourd'hui, l'insécurité juridique est préjudiciable à tous, et d'abord aux acteurs de l'éducation : enseignants, chefs d'établissement et directeurs d'école. Malgré la légalité de ces circulaires qui n'ont jamais été abrogées, leur interprétation a varié au gré des déclarations contradictoires de certains ministres. Il revient par conséquent au législateur de lever les contradictions qui persistent, de clarifier la question, et de régler une situation qui aurait dû l'être depuis longtemps, avant qu'elle ne devienne explosive et ne soit instrumentalisée par les extrêmes.

invité le législateur à clarifier la question que nous examinons aujourd'hui. En vain ! S'appuyant sur un arrêt de 1941, il soulignait que, entre l'agent et l'usager, la loi et la jurisprudence n'ont pas identifié de troisième catégorie de collaborateurs ou participants, qui serait soumise en tant que telle à l'exigence de neutralité religieuse En 2014, le Conseil d'État a confirmé la spécificité du service public de l'éducation dans son dossier thématique sur le juge administratif et l'expression des convictions religieuses, l'exemple le plus significatif étant celui de la loi du 15 mars 2004 qui impose, à juste titre, une neutralité aux usagers directs du service public de l'éducation, c'est-à-dire les élèves, dans le but premier de les protéger contre toute forme de prosélytisme, à un âge où l'individu se construit. Elle leur interdit de manifester ostensiblement leur appartenance religieuse pendant le temps pédagogique. Néanmoins, le Conseil d'État souligne qu'il reste paradoxalement possible pour les accompagnants des sorties scolaires de manifester leur appartenance religieuse. Il nous faut lever cette contradiction, car les activités pratiquées à l'occasion d'une sortie viennent nécessairement en appui des programmes et s'intègrent au projet au projet pédagogique de la classe, comme l'indique la circulaire de septembre 1999. Pour parvenir à la clarification attendue, il nous faut nous attarder à la fois sur le principe de neutralité et sur la nature de toute sortie scolaire, tout en rappelant quelques évidences. La notion de neutralité dans le service public de l'éducation nationale s'est construite au fil du temps par la loi et la jurisprudence, et ce depuis Jules Ferry : neutralité des agents, des enseignants et des usagers.

que, quelle que soit la qualité en laquelle elles interviennent, les personnes qui, à l'intérieur des locaux scolaires, participent à des activités assimilables à celles des personnels enseignants, soient astreintes aux mêmes exigences de neutralité. La sortie scolaire, quant à elle, est une activité qui prolonge l'enseignement en classe hors les murs de l'établissement. Elle intervient sur le temps scolaire obligatoire pour l'élève. Elle est organisée par l'enseignant dans un but pédagogique et ne constitue pas une activité de loisir extrascolaire. À ce titre, elle représente bien un prolongement du service public de l'éducation. Sa neutralité, quelle qu'en soit d'ailleurs la nature, doit donc être respectée. La sortie scolaire repose de son côté sur le volontariat des accompagnants, qui répondent à une sollicitation de l'enseignant. Cette démarche volontaire n'a pas vocation à se transformer en un droit.

classe. Il peut même arriver qu'il participe à la pédagogie de l'activité avec le professeur. Ce sont autant d'éléments qui fondent la nature juridique de l'accompagnant et qui démontrent que la sortie scolaire s'inscrit dans le prolongement de la mission de service public de l'éducation. Le texte de la commission, à la suite des nombreuses auditions de notre rapporteur Max Brisson, que je remercie pour son travail, me paraît satisfaisant en ce qu'il soumet les personnels de l'éducation et toute personne participant au service public de l'éducation aux mêmes valeurs, dont la liberté de conscience et la laïcité. Sa traduction juridique, par l'extension claire et sans ambiguïté du champ d'application de la loi du 15 mars 2004, me paraît de nature à offrir une solution aux problèmes rencontrés par le corps enseignant. Les membres de mon groupe se prononceront individuellement, en conscience, sur ce texte. Quant à moi, estimant que l'on ne peut pas laisser les directrices et directeurs d'école dans l'insécurité juridique, et suivant mes convictions, je voterai en faveur de ce texte. La parole est à M. Antoine

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici réunis dans cet hémicycle quelques jours seulement après l'outrance prétendue laïque d'un élu du Rassemblement national, plus soucieux d'agiter le peuple avant de s'en servir que de respecter le droit et les libertés de ses concitoyens. L'acte discriminatoire passé et la réalité du droit posé, il eût été sage que celui-ci présente publiquement ses excuses. Au lieu de cela, nous avons eu droit aux débats malsains, aux amalgames scandaleux et à un déversoir de haine. Cette polémique ne vise qu'un seul objectif : faire le lit de tous les extrêmes. On ne peut donc que regretter que, en dépit d'un contexte malaisé, le présent débat soit maintenu. Je l'ai dit en commission et le redis ici : ne pas céder à la provocation est aussi un acte républicain Avant d'entrer dans le détail, je dois avouer l'étonnement qui a été le mien quand j'ai vu ce texte proposé par la droite sénatoriale, la même droite qui s'était vivement opposée, il y a deux ans de cela, à l'un de mes amendements tendant à mettre fin à la rémunération des prêtres par la collectivité territoriale Vous en conviendrez, mes chers collègues, notre passion commune pour la laïcité peut décidément avoir des priorités surprenantes. Monsieur le ministre, vous avez rappelé avec justesse les principes qui régissent la laïcité de notre République. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire, mais aussi l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient nos croyances ou nos convictions. C'est aussi la stricte neutralité de l'État à l'égard du fait religieux. Dans le milieu scolaire, un vade-mecum rappelle avec clarté le cadre de cette neutralité. Aujourd'hui, aucune loi n'interdit à un adulte qui accompagne une sortie scolaire de porter un signe ostensible de religion, sauf en cas de prosélytisme. En effet, la neutralité religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées s'applique seulement aux enseignants, aux employés de la fonction publique et aux élèves. L'objectif annoncé par les auteurs de ce texte est de clarifier la situation. loi crée une nouvelle catégorie de personnes qui « participent » au service public de l'éducation. Or l'étude du Conseil d'État de 2013 affirme que le parent d'élève demeure un usager du service public, y compris lorsqu'il accompagne une sortie scolaire. En effet, le caractère bénévole de la tâche confiée aux parents accompagnateurs ne permet pas, à mon sens, de les assimiler à des collaborateurs occasionnels. En revanche, il revient aux chefs d'établissement de prévenir, voire de signaler tout acte prosélyte qui constituerait un trouble à l'ordre public et au bon fonctionnement du service public. L'état actuel du droit, que certains jugent ambigu, révèle en fait l'équilibre lumineux trouvé par la loi et la jurisprudence pour concilier les principes si exigeants qui fondent la laïcité. Ce silence sur les signes religieux, Aristide Briand, rapporteur de la loi de 1905, l'explique mieux que je ne pourrais le faire : « Le Le silence du projet de loi n'a pas été le résultat d'une omission. [ ...] Il a paru à la commission que ce serait encourir [ ...] le reproche d'intolérance et même s'exposer à un danger plus grave encore, le ridicule, que de vouloir, par une loi qui se donne pour but d'instaurer dans ce pays un régime de liberté, [ ...] imposer de modifier la coupe de [ses] vêtements. » Ainsi, une fois l'État et les Églises séparés, la kippa, le foulard, la croix ou le turban deviennent des accessoires et des vêtements comme les autres, portés par qui le souhaite. Une fois cela dit, la loi peut toujours évoluer, mais doit-elle régler les convictions intimes qu'elle suppose chez les adultes ? Le pourrait-elle seulement ? Mes chers collègues, les évolutions du paysage religieux ne doivent pas nous conduire à remettre en cause l'esprit de la loi de 1905. Je crois qu'il nous faut au contraire prendre appui sur ses piliers : la liberté de croire, la neutralité et le non-subventionnement des cultes pour apporter des réponses pragmatiques aux questions nouvelles. ce bel usage qui veut que les enseignants sollicitent des parents pour participer à l'encadrement d'une sortie scolaire s'organise déjà dans le cadre d'un dialogue, d'une relation de confiance entre l'école et ces parents. Dans cet échange, les enseignants rappellent le cadre laïque de l'école et peuvent inviter les parents à s'y conformer, sans pour autant les y obliger. De même, il faut le dire, le port d'un signe religieux lors d'une sortie est moins un droit exercé par les parents qu'une tolérance dans le pacte de confiance qu'ils nouent avec l'école. À cet égard, la récente affiche revendicatrice de la FCPE me semble tout aussi contre-productive et inadaptée que la présente proposition de loi. Nous le savons, dans certaines écoles, l'interdiction du foulard- disons-le, puisque c'est de cela qu'il s'agit -placerait les enseignants dans des situations inextricables au détriment des élèves. Plus grave encore, elle pourrait éloigner certains enfants de l'école publique, lorsque notre priorité commune est justement de ramener tous nos concitoyens vers la République. Mes chers collègues, ne cédons pas à la tentation de faire de la laïcité un territoire guerrier sur lequel nous lutterions contre le communautarisme. En la matière, notre assemblée a su, sur l'initiative de notre collègue Françoise Gatel, apporter une réponse législative adaptée pour mieux contrôler les écoles hors contrat. Nous devons aussi travailler à des solutions efficaces pour lutter contre la déscolarisation et mieux contrôler l'enseignement à domicile. J'entends parler ici de courage de légiférer. Mais le véritable courage ne serait-il pas d'assumer le principe selon lequel la liberté doit être la règle et la restriction de police, l'exception ? La laïcité léguée par les législateurs de 1905 n'est ni un glaive ni un bouclier. Elle est le cadre au sein duquel il nous faut élaborer les réponses pragmatiques qui, sans être simples, permettent de préserver le vivre ensemble de notre société. de notre société. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, c'est parce que nous jugeons cette proposition de loi inutile et inadaptée que notre groupe s'y opposera avec fermeté ! La parole

Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut une réponse globale aux dérives communautaristes. À l'évidence, dans ce domaine, le port du voile est un élément emblématique, car, dans certains quartiers, il prend une telle ampleur que l'on en vient à se demander si l'on est encore en France Or, si nous en sommes arrivés là, c'est aussi le résultat d'un certain laxisme généralisé depuis des décennies. Dans le passé, tout le monde savait qu'il existait un problème lié au port du voile chez les accompagnateurs de voyages scolaires.

? Pire encore, au niveau local, certains responsables politiques soutiennent les dérives communautaristes dans un but purement électoraliste. À juste titre, l'actuel ministre de l'intérieur s'est lui-même inquiété de ce qu'il appelle des « Molenbeek à la française », c'est-à-dire des villes où le communautarisme s'épanouit avec le soutien de la municipalité ou des élus locaux. On en trouve partout : ainsi, dans mon département, un maire s'est vanté de gagner les suffrages des musulmans en étant le seul en France à avoir financé avec 100 % de fonds publics la construction d'une mosquée. C'est interdit ! Non, c'est autorisé en Alsace-Lorraine,

et même l'installation de lampadaires décorés du croissant islamique dans la rue qui donne accès à la mosquée ! Ça suffit ! Alors, faut-il s'étonner

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les dispositions dont nous discutons aujourd'hui ont déjà été votées par le Sénat lors des débats sur la loi dite « pour une école de la confiance des travaux de la commission mixte paritaire, votre majorité a choisi de ne pas les retenir. Elle a accepté cette « concession mineure » selon l'expression du rapporteur, parce que le dispositif d'un autre amendement a été intégralement repris dans la loi définitive.

dans les écoles publiques et les établissements publics locaux d'enseignement, à leurs abords immédiats et pendant toute activité liée à l'enseignement. » Voilà ce que vous avez voté ! C'est excellent ! La portée de cette interdiction est bien plus large que celle dont nous débattons aujourd'hui. On peut donc légitimement se demander pourquoi vous avez déposé, moins d'une semaine après l'adoption définitive de la loi par le Sénat, une proposition de loi qui reprend une une mesure rejetée par la commission mixte paritaire au profit d'un dispositif plus général d'application directe. Les polémiques suscitées, initiées ou provoquées par cette proposition de loi éclairent sans conteste son objet essentiel. L'intention n'est pas de discuter de nouveau de la loi dite « pour une école de la confiance » que vous avez adoptée. Déposé cinq jours après l'adoption définitive de la loi par le Sénat, ce texte sert de prétexte à un débat sur la place du voile dans notre société. Elle nourrit la suspicion plus générale selon laquelle certains de nos concitoyens, par leur origine familiale, leur religion ou leur tradition, ne pourraient pleinement appartenir à la Nation, qu'il y aurait des dispositions religieuses fondamentalement incompatibles avec la citoyenneté républicaine. Eh oui ! Un lien de causalité pourrait même être établi entre une pratique religieuse d'ordre vestimentaire, la volonté de créer au sein de la République des communautés souhaitant échapper à ses lois et ce qu'Amin Maalouf appelle très justement les « identités meurtrières » qui se construisent dans la haine d'autrui. Cet amalgame n'est pas acceptable Puisque le débat porte finalement sur la fonction politique de la laïcité dans notre société, j'aimerais rappeler ici que celle-ci a été introduite dans la Constitution de 1946 par un amendement déposé par notre collègue et député communiste Étienne Fajon. à l'article premier de cette Constitution, « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Cet article fut complété dans la Constitution de 1958 par les deux phrases suivantes : « Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » L'essentiel est dit et la force de ces principes constitutionnels devrait nous inciter à plus de retenue, de circonspection et de sagesse, dès que l'on tente de les corriger pour en atténuer la portée Défendre la République, c'est aussi protéger celles et ceux que l'on veut rejeter hors de la Nation en raison de leurs origines ou de leurs croyances. Cette ardente obligation de l'État de défendre tous nos concitoyens victimes du racisme s'impose encore avec plus de force depuis l'attentat perpétré hier contre la mosquée de Bayonne. La laïcité ne peut être l'instrument de l'exclusion elle est au contraire le principe qui, en imposant la neutralité de l'État, permet l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de naissance ni de religion. D'aucuns appellent, y compris dans cette assemblée, à l'avènement d'une « nouvelle » laïcité, d'une laïcité « intégrale ». Ce surcroît de rigorisme obligerait les élus à une stricte neutralité religieuse par exemple, alors que, jadis, le chanoine et député Félix Kir montait à la tribune en soutane. Dans le même esprit, la neutralité religieuse qui s'impose aujourd'hui à tous les agents du service public devrait aussi s'étendre à tous les services pour le public, même privés. Un débat sur ces thèmes est légitime. Mais il mérite mieux qu'une discussion sur une proposition de loi de circonstance de deux articles, reprenant des dispositions déjà écartées. En ce qui nous concerne, nous sommes disponibles pour travailler sur ces sujets. Nous le sommes d'autant plus que notre histoire nous porte à défendre une laïcité au service de l'émancipation intellectuelle, politique et sociale. Monsieur le rapporteur, vous avez cité à plusieurs reprises Jean Zay, le ministre du Front populaire assassiné par la Milice. Comme vous, nous partageons son idéal, son programme et son action politique en faveur de l'éducation nationale.

d'une école « sans Dieu ». En septembre 1939, alors que le ministre de l'intérieur Albert Sarraut demandait le renvoi hors de France des enfants des réfugiés républicains espagnols, Jean Zay affirma seul, avec force, notre devoir moral de les maintenir dans les classes, au nom de la mission humaniste et universaliste de l'école. C'est toujours notre source d'inspiration, et c'est pourquoi nous voterons contre ce texte

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme dans tout débat, il est important de savoir de quoi l'on parle. Aujourd'hui, la proposition de loi qui nous est présentée- je m'interroge d'ailleurs sur son opportunité, à l'heure où les polémiques enflamment le débat public -concerne le port du foulard des mamans accompagnatrices de sorties scolaires, et rien d'autre Je suis convaincue par ces mots : « laïcité de l'État, pas de la société ». Cela veut dire trois choses. D'abord, cette expression signifie que la France garantit la liberté de conscience et de pratique, lorsque cette pratique s'inscrit dans la tolérance et le respect des valeurs républicaines. Enseignante, j'ai exercé dans un collège en zone d'éducation prioritaire à Melun, en Seine-et-Marne, où j'ai également été adjointe au maire pendant trente Je connais bien ces femmes qui, pour la plupart, vivent dans des quartiers difficiles. Il est caricatural de penser que la totalité de ces Françaises musulmanes utilisent le foulard comme l'étendard d'un projet islamique. Plus simplement, elles veulent vivre dans une société ouverte, tolérante, respectueuse de toutes les religions, en préservant des traditions familiales. Si l'on interdit à ces mamans d'accompagner leurs enfants lors de déplacements scolaires,

Interdire le port du voile risque, à l'opposé de l'objectif visé, de compromettre leur intégration sociale. En les stigmatisant, on les enferme dans leurs pratiques, on renforce le communautarisme, on empêche, paradoxalement, l'islam d'évoluer avec la société. L'école est parfois le seul lieu de socialisation pour ces femmes. laïcité de l'État, pas de la société » signifie aussi que l'État n'a pas à se plier aux revendications communautaires. Il doit veiller à lutter contre une certaine vision de l'islam incompatible avec les valeurs de la République, sans céder aux pressions électorales, aux caricatures et sans faire de concessions. Il doit également veiller à apaiser les tensions entre communautés, en s'opposant avec la plus grande fermeté à toute démonstration de haine à l'encontre d'une communauté ou d'une autre. Enfin, ces quelques mots veulent dire que nous devons, collectivement, veiller à ce qu'aucun enfant ne soit victime de prosélytisme dans le cadre de l'école publique, publique, à ce qu'aucune pression d'ordre religieux, même insidieuse, ne porte atteinte à la liberté de conscience de l'enfant, par définition vulnérable et influençable. Fions-nous à l'intelligence des enseignants, des directeurs d'établissements et, en dernier ressort, au juge pour garantir l'application éclairée du principe de laïcité. La réponse au communautarisme n'est pas la stigmatisation qui exacerbe les tensions. L'école, à mon sens, doit rester un sanctuaire, un abri pour permettre à tous les enfants de grandir avec les valeurs républicaines. Mais la France n'a jamais prôné l'égalitarisme. Elle ne saurait écarter une communauté qui lui paraît étrangère, mais, finalement, reflète une partie d'elle-même. Vivre en démocratie, c'est accepter les différences culturelles et religieuses de chacun de ses membres. Dès la petite enfance, c'est trouver la paix et l'entente, par-delà les différences. Pour autant, cette tolérance n'est pas sans limites, nous le savons, comme l'interdiction du voile intégral l'a démontré en 2010, comme l'obligation de neutralité religieuse à l'école l'a démontré en 2004, comme le renforcement du contrôle des écoles coraniques et des enfants déscolarisés l'a démontré encore récemment. D'autres lois viendront probablement, des lois que j'estime nécessaires, sur la formation et le contrôle des imams, sur le mode de financement des mosquées, sur l'évolution de notre système d'intégration. Les questions soulevées par ce débat sont éminemment plus complexes, plus vastes, que la réponse qui nous est proposée à travers ce texte. Il me semble que la réponse la plus saine pour désamorcer ces tensions consiste à réaffirmer, au sein de la République une et indivisible qui est la nôtre, les principes de tolérance, de liberté de conscience, de fraternité entre les communautés, et de partage des valeurs républicaines. Je pense que le respect de nos différences s'enseigne dès le plus jeune âge, par la confrontation aux autres, par le dialogue et l'ouverture. Ce que nous devons vraiment combattre, ce n'est pas le port du voile par quelques femmes qui démontrent, en participant à des sorties scolaires, leur implication dans l'éducation de leurs enfants. Ce que nous devons combattre, c'est le glissement d'une partie des musulmans vers une pratique radicale de l'islam ; c'est l'obscurantisme religieux, les haines communautaires et l'aliénation des femmes. Nous connaissons tous cette mère exemplaire meurtrie dans sa chair après l'assassinat de son fils par le terroriste Mohammed Merah. Depuis 2012, Latifa Ibn Ziaten, au sein de son association IMAD pour la jeunesse et la paix, circule dans les établissements scolaires pour venir en aide aux jeunes des quartiers en difficulté. Il faut conclure. Elle porte le voile sans que cela pose problème. Pour finir, je tiens à préciser que je m'exprime à titre personnel, et au nom de plusieurs des membres de mon groupe Les Indépendants - République et Territoires, mais chacun aura sa liberté de conscience

mais il est plus difficile de voir ce que l'on voit -, par manque de courage, ce sont hélas les extrémistes de tous bords qui se sont emparés, non pas du débat, mais des failles dans les lois de notre République.

Je tiens d'ailleurs à votre disposition, monsieur le ministre, une proposition de loi de même teneur pour les universités. Du respect de la neutralité religieuse à l'école, certains n'ont voulu voir qu'un prétexte de racisme, voire de « haine contre les musulmans Mais nous sommes en vérité bien en dessous d'Atatürk ! Le sujet n'est pas du tout celui-là ; il est celui du risque de fracturation profonde de notre pays, laïque et républicain, et, au premier rang, de son école publique. Voulons-nous abandonner notre modèle pour l'enseignement laïque, issu des lois de Jules Ferry et des décrets de Jean Zay ? Voulons-nous abandonner le creuset de l'école républicaine, sans distinction de race, de sexe et, à la suite de Portalis, de religion ? Voulons-nous abandonner les combats des féministes, chère Laurence Rossignol ?

! Si cela devait être, préparons-nous à vivre, selon une expression redoutable de l'ancien ministre chargé des cultes, plutôt « face à face » que « côte à côte Préparons-nous aussi à modifier l'article 1 de notre Constitution sur l'unité et l'indivisibilité de notre République. Sans texte clair, sans cadre légal, les positions des uns et des autres seront inconciliables : là est le risque grave de fracture de la République ! Voilà pourquoi,

Robert Badinter nous l'a dit, lui qui sans nul doute aura sa médaille sur nos travées : « Ce qui n'est pas illégal n'est pas forcément bienvenu. » Selon lui, le voile ne marque pas une « bonne volonté de vivre ensemble », étant rappelé que le port du voile n'est pas une prescription canonique.

lors, mes chers collègues, sans distinction de sensibilité, nous ne devons pas abdiquer. Quel courage ! Nous ne le devons pas, pour être dignes des Lumières et des pères de la République, Jules Ferry- notre prédécesseur en ces lieux Nous ne le devons pas pour l'école, mais aussi pour tous les croyants, tous les agnostiques et tous les athées de France qui se retrouvent dans cette école de la République.

Face aux extrémistes, nous ne pouvons pas avoir la main tremblante ! Je vous demande donc, très solennellement, de soutenir sans réserve ce texte sur la laïcité, qui porte le sceau, selon les mots du Général, de l'honneur, du bon sens, de l'intérêt supérieur de la patrie.

Ce qui est en question, dans cette affaire, c'est la remise en cause régulière des valeurs de notre société et de notre vivre ensemble par les tenants d'une vision de l'islam communautariste et radicale. Nous en sommes là aujourd'hui, car, depuis plus de vingt ans, les gouvernements successifs ont manqué de lucidité, ont fait preuve de lâcheté et n'ont pas eu le courage ni de gérer l'immigration ... Il y a un lien ! ... ni d'adopter une ligne politique claire. Cette ambiguïté a alimenté les tensions, attisées par les tenants d'un islam politique qui tente de remettre en cause notre société et ses valeurs républicaines. Les sorties scolaires, puisque c'est bien d'elles qu'il s'agit, sont effectuées dans le cadre du temps scolaire et, à ce titre, doivent être soumises aux règles régissant l'obligation de neutralité des agents publics, indépendamment des fonctions exercées. Ainsi, lorsque des parents se portent volontaires pour accompagner une sortie d'élèves, ils deviennent eux aussi, même bénévoles, des collaborateurs occasionnels du service public. Il serait donc logique que les sorties soient considérées comme partie intégrante du temps scolaire et de l'environnement scolaire, et que les règles de neutralité vestimentaire soient appliquées dans ce cadre, comme à l'intérieur de l'établissement, pour toutes les personnes concourant à encadrer et éduquer les enfants. L'école est le reflet de notre société ; c'est aussi le lieu où la France de demain se construit. Ce n'est pas avec de belles citations, de jolies petites phrases que le problème Le communautarisme est en train de ronger la société française, il la fracture, la divise, créant des tensions de plus en plus vives. Il suffit de lire, l'excellent ouvrage du politologue politologue Jérôme Fourquet, pour comprendre le glissement sociétal que nous vivons. Nous avons été incapables d'intégrer ou de combattre les ghettos : nous en subissons aujourd'hui les effets mes chers collègues, que je me focalise uniquement sur les signes extérieurs de la religion islamique, je vous dirai la même chose s'il s'agissait d'accompagnateurs coiffés d'une kippa ou d'un turban, ou d'accompagnatrices vêtues d'une robe bouddhiste. Arrêtons de nous cacher derrière la bien-pensance ! Aujourd'hui, ce sont les maires et les directeurs d'école qui gèrent seuls, tant bien que mal, ces questions au quotidien, en composant avec le flou entretenu en haut lieu depuis de trop nombreuses années. nous parlons aujourd'hui du voile, mais que dire du prosélytisme de certains animateurs, des revendications sur les menus des cantines scolaires ou pour l'obtention d'horaires spécifiques pour les femmes à la piscine Notre Constitution de 1958 dit que « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Puisqu'il n'y a plus de religion d'État dans notre pays, la religion doit s'exercer uniquement dans un cadre privé et ne doit en aucun cas influencer d'une façon ou d'une autre l'opinion des enfants, qui se forment, sur le temps scolaire, dans un cadre strictement laïque. A-t-on jamais forcé un parent d'élève à accompagner une sortie scolaire ? Si, pour une mère de famille, retirer son voile et montrer ses cheveux est insupportable, elle peut rester chez elle, mais qu'elle ne prétende pas collaborer à un service public laïque et démocratique sans en accepter les règles. Car il faut être lucide, c'est un véritable bras de fer qui est engagé par ces femmes brandissant le voile comme un étendard, appuyées par un communautarisme islamiste, politique, qui s'est fixé pour objectif d'utiliser chaque faille dans notre État de droit pour y imposer sa morale religieuse, faisant peu à peu de notre pays, non plus une Nation, mais un pays avec des communautés vivant les unes à côté des autres. Il est temps de choisir quel modèle de société nous souhaitons : vivre ensemble ou vivre à côté les uns des autres Le Gouvernement nous dit : « On n'y peut rien, c'est la loi. » Mais la loi est faite pour évoluer ! Elle est faite pour s'adapter aux changements de la société, et nous autres parlementaires sommes là pour accompagner cette évolution ! Pour cela, il faut du courage. Il faut, pour une fois, avoir le courage d'entendre ce que disent les Français et comprendre ceux qui voient leur quartier et leur commune s'enfoncer peu à peu dans le communautarisme, leur environnement se transformer et les propos se radicaliser. J'ai entendu récemment dans un débat : « Il suffit de généraliser la viande halal. Comme ça, tout le monde pourra en manger ! » Pourquoi ne pas imposer de manger casher dans ce cas ? Personnellement, je préfère manger du poisson le vendredi ! Mais au nom de quel principe devrait-on soumettre le droit commun et la pratique commune au caprice des religions, dans une République laïque et indivisible ? Moi, j'ose encore croire en la France ! Je crois aux valeurs de notre République et je me refuse à les voir grignotées insidieusement par des idéologies politiques, radicales et communautaristes, mettant à mal nos valeurs communes et notre vivre ensemble.

me paraît délicat et un peu perdu d'avance ! Mais je voudrais partager avec vous un sentiment et quelques réflexions. Mon sentiment, c'est celui- extrêmement désagréable -d'être prise dans un étau. La première mâchoire de cet étau est celle de la haine et du racisme, celle qui déteste les musulmans comme elle a toujours détesté les Arabes, celle qui n'a jamais été laïque, celle qui n'a jamais autant aimé la France que quand elle n'était pas la France. J'invite mes collègues de la droite républicaine à ne pas s'émouvoir quand je parle de l'extrême droite. Je ne parlais pas de vous jusqu'à présent,

est celle de l'extension de l'emprise religieuse dans la société française, notamment de l'islam politique. En effet, autant la foi est un sujet intime, autant la religion est une question politique. La première étape stratégique des doctrinaires passe par la réislamisation des musulmans de France. Il s'agit de communautariser les musulmans autour du fait religieux dans l'espace public, en opposant progressivement une pratique religieuse de plus en plus rigoriste à la laïcité républicaine. Pour ceux-là, aussi, le port du voile est l'objet symbolique de leur visibilité, même si, paradoxalement, cette visibilité passe par l'invisibilité des femmes. Les uns comme les autres ont donc objectivement intérêt à installer le voile au centre du débat public. Bien sûr ! Pour les promoteurs de l'islam politique, plus on parle du voile, de sa place et de sa compatibilité avec la République, mieux c'est, car c'est avec ce drapeau qu'ils comptent bien susciter la solidarité communautaire. Si le voile devient un objet de racisme, alors il devient aussi le signe de la résistance au racisme, et c'est le pire des scénarios C'est le scénario de l'escalade : d'un côté, Dijon et son conseiller régional haineux, indigne, qui la nourrit ; de l'autre, la coalition des naïfs qui laissent prospérer l'islam politique, abandonnent celles et ceux qui résistent et choisissent le confort moral du déni. Et nous, mes chers sur une ligne de crête, pesant chacun de nos mots, chacun de nos actes, pour ne renforcer ni un camp ni l'autre. Certains diront que c'est pleutre. Je me contenterai de dire que c'est précautionneux. Il faut agir dans le bon ordre. À mes yeux, réduire la fracture qui s'est installée dans notre société est le préalable à toute reconquête républicaine. Cette proposition de loi n'y contribuera pas. Je crains même qu'elle ne soit, si j'ose dire, du pain bénit pour les islamistes, une occasion supplémentaire de coaliser et de communautariser les musulmans, y compris ceux qui n'ont pas cette pratique rigoriste de l'islam. Très bien ! Je ne pense pas non plus que cette proposition de loi rendra la laïcité plus aimable ou plus désirable à qui que ce soit. Défendre la laïcité, c'est en faire un usage juste et constant. La laïcité, ce n'est pas exalter à tout propos l'identité chrétienne de la France ou convoquer les évêques à tout bout de champ pour solliciter leur avis sur le droit des femmes à disposer de leur corps ! La laïcité, c'est un projet de société, qui suppose la justice et l'égalité.

Ce que nous payons aujourd'hui, c'est l'abandon des quartiers populaires, l'absence de perspective pour ceux qui y vivent, la ségrégation spatiale et notre inefficacité à lutter contre le racisme. Tant qu'un jeune avec un prénom musulman aura cinq fois moins de chances de trouver un travail qu'un jeune avec prénom d'origine catholique, ... Ce n'est pas vrai ! ... il ne sera pas possible de convaincre ce jeune que la République et l'égalité sont faites pour lui et à partager avec lui ! Quand le relief est incertain, quand le paysage est trouble, il faut une boussole. La mienne tient en trois questions. Avec cette proposition de loi, allons-nous réduire la fracture qui s'est installée entre les Français ? Allons-nous désarmer les haineux de tous bords ? Allons-nous nous extraire du face-à-face sinistre entre les identitaires des deux camps ?

la France est une République laïque. Cette règle, fruit de notre histoire, a longtemps divisé notre nation, mais, aujourd'hui, elle la rassemble et elle doit la rassembler La laïcité n'est pas seulement un droit ; c'est un devoir ! Elle exige d'accepter des règles communes, indispensables à l'équilibre de la société, au premier rang desquelles la neutralité des services publics. Le législateur a voulu faire de l'école un espace neutre d'un point de vue religieux, pour permettre à l'élève de se construire librement en tant que citoyen, en le protégeant contre les influences et les passions extérieures. Cette conquête d'une école laïque s'est faite par étapes. Il y a d'abord eu la substitution à l'enseignement d'une morale religieuse d'une instruction morale civique et laïque, puis la suppression en 2004 des signes ostensibles d'appartenance religieuse dans les établissements scolaires. Il faut aujourd'hui franchir une nouvelle étape en inscrivant dans la loi le principe de neutralité religieuse applicable à toute personne participant aux sorties scolaires, ce qui est déjà le cas pour les enfants et les enseignants, mais pas pour les accompagnants. Il est donc temps de mettre fin à cette incohérence juridique Je ne comprends pas la posture de désintérêt du Président de la République, qui affirme que le port du voile dans l'espace public n'est pas son affaire. Doit-on lui rappeler que les sorties scolaires sont des temps pédagogiques s'inscrivant dans le temps de l'éducation nationale ? Cela fait bien longtemps que l'enseignement scolaire ne se limite plus aux quatre murs de la classe. Cette ouverture vers l'extérieur nous invite à repenser le principe de laïcité appliqué à l'école. Chaque sortie nourrit un projet pédagogique et fait l'objet d'une préparation en amont. Il n'est donc pas possible de déconnecter les enseignements scolaires en classe de ceux qui sont dispensés à l'extérieur. La sortie scolaire n'est en réalité qu'un prolongement des enseignements délivrés en classe, une école « hors les murs La neutralité religieuse doit donc aussi s'y appliquer, de la même façon qu'elle s'applique en classe, de la même façon qu'elle s'applique dans le gymnase ou la salle municipale accueillant les activités d'éducation sportive. Cette proposition de loi est également la suite logique des récentes évolutions jurisprudentielles, qui tendent vers toujours plus de neutralité des parents d'élèves. En juillet dernier, la cour administrative d'appel de Lyon a admis la légalité d'un règlement intérieur imposant la neutralité religieuse à toute personne, y compris les parents d'élèves, intervenant dans une classe pour participer à des activités assimilables à celles des enseignants. Par ailleurs, si le Conseil d'État estime que les parents d'élèves ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité religieuse, il a toutefois précisé que le chef d'établissement peut leur recommander de s'abstenir de manifester leur appartenance ou leur croyance religieuses. Cette situation entraîne des décisions différentes d'un établissement scolaire à l'autre, au grand dam des parents d'élèves et des élus locaux. Le droit actuel et l'ambivalence du Gouvernement sont sources de polémiques et de tensions, comme l'ont récemment montré les affiches de campagne de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves, défendant le droit pour les mères voilées de participer à des sorties scolaires. Monsieur le ministre, alors que plusieurs de vos collègues ont multiplié les prises de position contradictoires- ce sont les limites du « en même temps » -, votre gouvernement doit sortir de l'ambiguïté. Les Français vous le demandent, puisque 66 % d'entre eux sont favorables à cette proposition de loi. Mes chers collègues, la laïcité que nous défendons n'est en aucun cas l'expression d'un sentiment antireligieux. C'est, au contraire, la liberté et la tolérance pour tous. Jacques Chirac affirmait en 2003 que le débat sur la laïcité renvoyait « à notre cohésion nationale, à notre aptitude à vivre ensemble, à notre capacité à nous réunir sur l'essentiel ». ans plus tard, la loi a juste besoin de clarté, et ce texte en apporte. Deux questions, mes chers collègues : la neutralité religieuse à l'école a-t-elle été pensée pour protéger les enfants ou les murs de l'établissement ? La sortie scolaire est-elle du temps scolaire ? La parole

l'importance des mots. Il est difficile d'être subtil et équilibré sur ces questions aujourd'hui : celui qui vous parle est bien placé pour le savoir. Lorsque j'ai dit « pas interdit, mais pas souhaitable », j'ai résumé l'état du droit actuel et j'ai résumé ce qu'ensuite Robert Badinter a dit. Il est bien normal que vous ayez plus de révérence pour les paroles de Robert Badinter que pour les miennes, mais en réalité ce sont les mêmes ! Exactement

qu'un accompagnant participe à une activité d'enseignement, et uniquement à une activité d'enseignement. Il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit- et, personnellement, je m'y refuse absolument ! En revanche,

N'est-il pas de bon sens que les personnes participant au service public de l'éducation, pour des activités liées à l'enseignement dans les établissements ou en dehors d'eux, soient également tenues de respecter ses valeurs, comme l'indique le texte de l'article 1 Dans notre société, de plus en plus fracturée par le fléau du repli communautariste, par les tentations du huis clos technologique ou de l'entre soi sociologique, « faire Nation » apparaît bien compliqué. Si « vivre ensemble » est devenu un slogan, c'est en fait désormais surtout un objectif, car ce n'est malheureusement plus une évidence. Or il est un lieu où l'on peut semer et faire germer les valeurs de la République, qui nous unissent ; un lieu où l'on transmet le savoir, où l'on ancre des valeurs, où les consciences se construisent, s'épanouissent et s'émancipent ; un lieu qui doit être protégé, préservé, sanctuarisé : c'est l'école de la République, véritable pré carré de la genèse citoyenne, libre et indépendante. Si c'est la République qui a instauré l'école moderne gratuite et obligatoire, c'est l'école qui a fortifié la République. Toutes deux sont indissociables, consubstantielles. Or, dès l'origine, cette école s'est voulue laïque, donc neutre, d'abord parce qu'elle entendait respecter tous ses enfants- ceux dont les parents croyaient au ciel ceux dont les parents n'y croyaient pas. Remercions d'ailleurs notre rapporteur pour ses rappels juridiques et historiques, précis et précieux : mieux vaut savoir d'où l'on vient pour ne pas se perdre. Le combat pour la laïcité a une histoire jalonnée de débats et de fièvres. On a évoqué les lois de 1882, de 1886 et de 1905 : personne aujourd'hui n'en conteste la légitimité ou l'utilité. On a aussi mentionné la loi de 2004, relative à l'interdiction du port de signes religieux ostentatoires par les élèves personne non plus ne la remet désormais en cause, bien au contraire. Or ce texte fut précédé de quinze ans de controverses et de polémiques nées, notamment, après l'affaire du collège Gabriel-Havez de Creil, dans le département de l'Oise, dont Jérôme Bascher et Laurence Rossignol sont, comme moi, les élus. vous serez surpris par leur actualité. À l'époque, certains refusaient la perspective de légiférer, sous prétexte de « stigmatisation ». On nous annonçait même que certains établissements scolaires allaient se vider de leurs élèves ! Il n'en a rien été : au contraire, cette loi a permis de retrouver un débat plus L'école admet toutes les fois, toutes les croyances, pour peu qu'on ne les montre pas. Il faut conclure. C'est valable pour les enseignants, pour les personnels administratifs et techniques et pour les élèves. Pourquoi ne le serait-ce pas pour les parents ? La parole est à M. Pierre Ouzoulias, sur l'article. Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous l'avez dit à plusieurs reprises : le voile n'est pas anodin. Sur ce sujet, je me permettrai de vous donner quelques éléments purement factuels, avec la double distance que me donnent mon statut d'historien et ma qualité d'athée- sans porter de jugement de valeur. Dans les trois religions du Livre, les religions juive, chrétienne et musulmane, le voile est la manifestation vestimentaire d'une position particulière de la femme au sein de la société. Tertullien,

Dans son travail d'histoire religieuse dédié au voile, Rosine Lambin montre que le christianisme est le premier monothéisme qui a construit la théorie religieuse de la morale de la coiffure féminine. Elle conclut ainsi : « Le voile Le voile des femmes est de souche méditerranéenne, donc à la fois occidental et oriental. [ ...] C'est l'occident chrétien qui a institué religieusement le voile. Je ne crois pas qu'il nous appartienne de légiférer en matière théologique ... Eh non ! ... et ce n'est pas à nous de décider ce que doit être la pratique religieuse des croyantes. En revanche, dans notre travail législatif, seules comptent les lois que nous nous donnons à nous-mêmes : il n'y a rien au-dessus qui puisse nous être imposé.

Il a fallu des siècles pour établir le Concordat, un siècle de plus pour séparer l'Église de l'État, puis pour affirmer ce concept de laïcité auquel nous sommes tous très attachés, j'en suis convaincu. On trouve bien quelques laïcards aigris qui voudraient pouvoir effacer totalement cette référence chrétienne, comme une sorte de revanche sur l'histoire. Chose étonnante, ce sont les mêmes qui militent pour ne porter aucune restriction à l'exercice d'autres cultes dans le domaine public. Rappelons que la religion musulmane n'oblige personne à porter en permanence un voile ou un foulard sur la tête. Ce bout de tissu est devenu un emblème politico-religieux pour ceux qui veulent défier la République, pour ceux qui veulent afficher comme une évidence la soumission de la femme. Ce bout de tissu, comme d'autres, est tout sauf insignifiant. Faut-il que nous soyons à ce point aveugles, face aux références historiques qui ont été rappelées, pour refuser d'encadrer tout ce qui concourt au service public ?

Alors, étendons à ces temps l'interdiction de signes ostensibles, dans le prolongement de la loi de 2004. Mes chers collègues, il y a une solution finalement assez simple au problème qui nous est soumis aujourd'hui demandons aux accompagnants de ces sorties scolaires d'enlever, pour quelques heures, ce bout de tissu. Cela ne les privera nullement d'exercer librement leur religion comme notre Constitution le leur garantit

de l'émergence d'une société de prohibition, d'interdiction et d'exclusion, qui ne fera que renforcer les extrêmes. On ne répond pas à une vision totalitaire de la société par l'instauration d'une intolérance institutionnelle vécue comme une humiliation.

d'invoquer la laïcité, comme le fait aujourd'hui une partie de la droite sénatoriale, ne laisse pas de m'interpeller : la même sensibilité politique s'est farouchement opposée au grand service public laïque et unifié de l'éducation nationale

Permettez-moi de m'étonner devant cette laïcité à géométrie variable : la laïcité ne se défend pas de manière occasionnelle ! L'unité de la Nation doit être notre préoccupation prioritaire, dans ces temps où les forces centrifuges minent notre modèle de société ; mais l'unité de la Nation ne peut être rabaissée à une uniformité mettant à mal ce que Jean-Paul Delevoye appelle très justement « le prosélytisme de l'empathie et de l'altérité

le calme dans nos établissements et dans nos assemblées de loi n'est pas le premier texte à s'en prendre aux mères accompagnatrices voilées. La droite va mal, son mauvais score aux élections européennes le confirme. En cette veille de municipales, elle cherche à mordre sur les plates-bandes de l'extrême droite, dans l'espoir de grappiller des voix.

alarmer la population ! D'ailleurs, selon un récent sondage, la lutte contre l'islamisme, souvent confondu avec l'islam, n'intéresserait que 56 % des Français, la santé et la lutte contre le chômage venant largement en tête. Voilà donc une droite faisant mine de lutter contre l'islamisme en enlevant leur voile aux mères accompagnatrices, quand d'autres, dignes héritiers de la vision paternaliste des colonisateurs d'antan, prétendent les émanciper des chaînes de l'oppression masculine musulmane. Marqueur identitaire pour beaucoup de femmes dans une France peinant à les intégrer, le voile est certes utilisé par des intégristes comme un signe de ralliement. Mais, heureusement, le libre arbitre est encore la la règle : 70 % des musulmanes y seraient favorables, ... Mais bien sûr ! ... sans avoir obligatoirement à le porter. Seule une laïcité inclusive nous mènera à l'intégration. La stigmatisation engendre le désordre en brisant la cohésion sociale. Occupons-nous plutôt des femmes battues et assassinées par leurs compagnons, de nos 9 millions de pauvres, ou encore du chômage, et luttons sérieusement contre la radicalisation avec un programme construit et de long terme !

Toutefois, il me semble déterminant que notre débat ne se focalise pas sur le port du voile, car il existe d'autres signes religieux susceptibles de provoquer des situations conflictuelles lors des sorties scolaires.

Imaginons qu'une accompagnante arrive vêtue d'un burkini : en l'absence d'une législation portant sur la neutralité religieuse, quelle sera la réaction des enseignants face au port de cette tenue, qui est un signe religieux manifeste ?

chroniquer dans la presse française tranquillement, alors qu'il a été condamné pour incitation à la haine religieuse et que le racisme est, non une opinion à débattre, mais un délit ; quand on est dans cette situation, on doit s'interroger sur l'opportunité des débats

sénatoriale, je vous pose la question : de quoi avez-vous peur ? Les valeurs de la République ne vous suffisent-elles plus ? Pourtant, la laïcité, c'est la liberté ; la laïcité, c'est l'égalité ; la laïcité, c'est la fraternité. La loi de 1905 assure ces valeurs, un point c'est tout. des mots prononcés par Aristide Briand avant le vote de la loi de 1905 : « La réforme que nous allons voter laissera le champ libre à l'activité républicaine pour la réalisation d'autres réformes essentielles.

Il faut donc toucher à ce sujet avec beaucoup de précaution ! Deuxièmement, on nous « bassine »- passez-moi l'expression ! -avec le service public de l'éducation nationale.

des écoles de la République française pour que leurs enfants puissent recevoir l'enseignement que la République leur doit ! Considérons-nous, encore

le département de la Réunion, où toutes les cultures, toutes les religions, coexistent de manière pacifique. On a pu y voir, voilà quelques semaines, l'évêque remettre les insignes de la Légion d'honneur à un imam,

a constaté, « à travers les réclamations reçues, que beaucoup d'incertitudes demeurent quant au champ d'application de ce principe de laïcité ». Il n'est donc pas illégitime de légiférer. Pour autant, j'ai du mal à comprendre la position du Conseil d'État, que vous avez fait vôtre, monsieur le ministre, au prix de quelques contorsions, lorsqu'il énonce que les parents ont le statut de simples « usagers », n'exercent pas une mission de service public de l'éducation

sauf à s'engager sur la voie des accommodements déraisonnables, de surcroît quand il s'agit de l'école, et à aller contre une partie de notre héritage républicain. C'est notre singularité, je crois, qui est précisément vilipendée parfois par les instances anglo-saxonnes qui, elles, ont fait le choix de reconnaître une forme de communautarisme. Or c'est l'honneur de notre histoire nationale que de faire de l'école un lieu sanctuarisé, dévolu à la transmission et protégé contre toute intrusion idéologique ou religieuse par le principe de neutralité religieuse. Je ne crois pas qu'il faille que notre pays s'aligne peu à peu, d'accommodement en accommodement, sur le modèle de sécularisation qui prévaut dans d'autres pays européens, c'est-à-dire sur la laïcité libérale qui, au nom d'une conception dévoyée de la tolérance, laisse une place aux influences religieuses, quelles qu'elles soient, dans les lieux ou dans le temps de l'école. L'école en dehors de l'école, à travers les sorties pédagogiques, c'est encore l'école Robert Badinter n'a pas dit autre chose sur la valeur de cette laïcité, qu'il a récemment qualifiée de « grande barrière contre le poison du fanatisme religieux ». Il a ajouté : « L'idée que l'on doit respecter l'autre signifie aussi que l'autre doit vous respecter. par conséquent de donner aux collaborateurs occasionnels du service public de l'éducation un statut spécifique, en fixant clairement leurs obligations et en tirant les conséquences de leur participation au temps pédagogique du point de vue du principe de neutralité, issu de notre laïcité.

d'abord eu la convention de l'extrême droite organisée par Marion Le Pen, Zemmour et compagnie, lesquels ciblent nos compatriotes musulmans comme un ennemi de l'intérieur. Puis l'agression verbale

Cette haine et ce rejet de l'autre renforcent la stigmatisation, le repli sur soi et le communautarisme. Il faut donc parler d'une voix claire et forte. Liberté, égalité, fraternité, tel est évidemment notre combat commun, mais c'est une autre question. À la société

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a quelques décennies, la question du port du voile par des femmes accompagnatrices lors de sorties scolaires ne se posait pas.

C'est pourquoi je voterai sans hésiter ce texte qui donne un cadre et aide les directeurs d'école, bien souvent pris entre le marteau et l'enclume, entre des parents qui se fâchent en voyant des femmes voilées et des femmes voilées qui insistent pour

La parole est à Mme Annick Billon, sur l'article. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, parce que j'estime qu'on ne doit pas laisser les directeurs seuls pour décider d'accepter ou non les signes ostentatoires lors des sorties scolaires, parce que j'estime que ces sorties effectuées sur le temps scolaire doivent respecter le principe de neutralité, parce qu'il

car elles refusent de porter le voile, et parce qu'aucune religion n'impose le port du voile, parce que parfois aussi- je dis bien : « parfois

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quelle est la fonction première de la loi ? Protéger les plus faibles, les plus fragiles ! Or dans notre société,

aujourd'hui, tous ceux qui ont contribué à bâtir le système de l'école publique laïque l'ont composé de cette façon.

je n'ai jamais hésité, j'ai toujours choisi l'enfant. Voilà pourquoi je voterai cette proposition de loi.

le vade-mecum de la laïcité et le Conseil des sages de la laïcité, de façon à nous adapter au cas par cas. Soyez assurés que ma consigne au quotidien, notamment vis-à-vis des inspecteurs de l'éducation nationale, est d'aider les directeurs d'école confrontés à cette situation. Encore une fois, ne généralisons pas ! Certaines situations

elle tend à accentuer la confusion juridique en étendant à davantage de personnes, d'une part, une interdiction et, d'autre part, l'obligation de respecter des valeurs. Le texte dont nous débattons aujourd'hui, sous couvert d'appliquer une laïcité sans concession, ne comblera aucun éventuel vide juridique. À l'inverse, il va complexifier l'état du droit tout en stigmatisant une catégorie de citoyens, des parents d'élèves et, par là même, leurs enfants. Nous ne sommes pas dupes quant au but de ce débat. En voulant étendre un article du code de l'éducation, issu de la loi de 2004, portant une interdiction destinée aux seuls élèves, qui- je le rappelle -sont des usagers particuliers du service public de l'éducation puisqu'ils sont soumis à l'obligation scolaire, le Sénat est en train de créer un amalgame entre deux catégories juridiquement distinctes les agents du service public, qui doivent respecter la plus stricte neutralité dans l'exercice de leurs fonctions, et les usagers, soumis à une simple obligation de discrétion liée à la nécessité du bon fonctionnement du service, auxquels la jurisprudence constante depuis 2013 a toujours assimilé les parents d'élèves, qu'accompagnateurs. En commission, le rapporteur a visé, de façon très large, toutes les personnes qui participent au service public de l'éducation et à tout moment ; le texte est ainsi potentiellement étendu aux intervenants extérieurs.

Le problème est que cette nouvelle catégorie n'est absolument pas définie par la loi et que ses contours juridiques pour le moins incertains ne manqueront pas d'entraîner des contentieux. Qui dit participants et obligations dit également droits et, éventuellement, traitements liés à la fonction de participant. Par

nous avons examiné cette proposition de loi et l'avons travaillée. La classe, c'est la classe dans les murs et hors les murs. Je ne vois pas pourquoi ce qui vaut pour la classe dans les murs ne vaudrait pas lorsque cette classe se déroule hors les murs, par exemple à l'occasion de la visite d'un musée.

qui a construit l'école publique dans les campagnes de France à la fin du XIXsiècle. Une laïcité accommodante n'aurait pas permis de construire la même école publique dans notre pays. On peut changer de position vis-à-vis de l'école, mais alors il faut l'assumer. En ce qui me concerne,

Au nom de la commission, je vous propose de ne pas supprimer cet article, et donc d'émettre un avis défavorable sur l'amendement, pour protéger ce bien précieux, cet héritage que nous devons aux pères fondateurs de l'école publique et qui fait toute la spécificité de l'école française. Cette école, il faut la protéger, et je vous propose de parachever le travail.

loi est absolument nécessaire. Je suis d'accord avec le ministre sur le fait qu'il y a voile et voile, que chaque situation est particulière et que le baromètre doit être le prosélytisme.

alors il faut l'exiger complètement. Par exemple, on ne peut pas continuer à convoquer au concert des nations respectables celles qui financent massivement dans tous les quartiers de notre pays, et dans plusieurs autres, l'islamisme politique,

vous nous avez expliqué à plusieurs reprises ici, dans cet hémicycle, que cette loi était une étape fondamentale, essentielle, pour faire progresser la laïcité et qu'elle était, par ailleurs, un moyen de

paritaire d'écarter cette disposition, si elle était aussi fondamentale que ce que vous nous présentez maintenant ? Par ailleurs, vous avez fait adopter, avec l'accord du Gouvernement, une disposition beaucoup plus large, beaucoup plus large, qui interdit toute forme de prosélytisme lié à l'enseignement. Expliquez-nous pourquoi, alors que vous avez fait voter cet amendement fort, vous nous dites maintenant qu'il est absolument inutile ? Vous vous répétez

comme je l'ai dit à propos de Tertullien, pourquoi ne l'interdisez-vous pas dans l'école privée ? Soyez logiques, allez jusqu'au bout de votre démarche laïque et féministe ! La parole est à M. Rachid Temal,

d'Aristide Briand : « La loi doit protéger la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dire la loi.

disait toujours : « On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. » Si, pour une fois, nous pouvions sortir de l'ambiguïté pour servir la République laïque, ce serait vraiment bien

Quand je dis « certains », je vise ceux qui, sur le terrain, essayent de faire avancer le communautarisme. Cette casuistique vous obligerait à faire une loi chaque fois qu'un vêtement vous paraîtrait bizarre ou chaque fois qu'on commencerait à trouver que quelque chose ne va pas. Dans les faits, cela est impossible et nous dévie d'ailleurs du but essentiel,

eu égard aux objectifs que vous affichez et que, par ailleurs, je peux partager.

dans le cadre d'activités liées à la classe. Avant la décision de la cour administrative d'appel de Lyon, ceux-ci pouvaient afficher leur croyance. Ils ne le peuvent plus

pour défendre l'école de la République, puisque l'école est bien le creuset de notre société et des valeurs dont nous ne cessons de parler. Cher Max Brisson, il y a longtemps que nous avons quitté l'école, nous nous sommes envolés et non pas « envoilés

pas celles et ceux qui la portent

Dans ce pays où des millions de catholiques pratiquent leur religion, les uns par conviction réelle, d'autres par habitude, par tradition de famille, il était impossible d'envisager une séparation qu'ils ne puissent accepter. Ce mot a paru extraordinaire à beaucoup de républicains qui se sont émus de nous voir préoccupés de rendre la loi acceptable.

la laïcité pour fracturer la société et créer des divisions. Je crois que nous devrions en rester à nos fondamentaux, demeurer inspirés par cette loi de liberté et ne pas en faire un carcan pour

C'est de réunir indistinctement les enfants de toutes les familles et de toutes les églises »- cela vaut aussi, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas dans les églises -« pour leur faire commencer la vie dans une atmosphère de paix, de confiance et de sérénité. » Je crois que, dans cet hémicycle, nous avons été à peu près

Monsieur le ministre,

Qu'est qu'une activité périscolaire ? C'est une activité qui se déroule à côté de l'enseignement traditionnel dispensé au sein des établissements.

héritage familial et vous fragilisez le message de l'école, qui permet justement de faire société en créant une distance entre l'enseignement scolaire

l'argument prétendument technique que vous employez n'en est pas un. Même si l'on s'en tenait à ce qu'a dit M. le rapporteur, à savoir qu'il ne s'agit que d'une qualification concernant les accompagnants, on ne réglerait pas le problème posé, car les parents d'élèves

indiquer explicitement la nécessité de s'abstenir de porter des signes ou des tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ou communautariste. C'est très important ! Je ne suis toujours pas convaincu par les propos tenus par M. le ministre de l'éducation nationale,

à Zora, Fatima, Leïla et Samia, ces élèves que j'ai eues jusque dans les années 2000, qui se sont battues pour sortir du carcan familial, de la pression des pères

J'espère que tous ceux qui s'apprêtent à voter le texte dont nous débattons ont bien à l'esprit que, en excluant des sorties scolaires les mères d'élèves portant un foulard, ce sont des classes entières que l'on va priver de sortie.

Je vais essayer de répondre à une intervention qui n'a pas eu lieu ... Les sorties scolaires sont du temps scolaire sur l'ensemble du territoire de notre République. pour que le texte soit appliqué à Wallis et Futuna, comme l'est la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux ostensibles pour les élèves, la loi doit expressément le prévoir. Pour ce qui concerne les autres territoires d'outre-mer, soit la loi

ne porte que sur l'affichage. Le prosélytisme, c'est un autre sujet ! Il s'agit ici de s'inscrire dans la logique d'une école publique où l'on n'affiche pas ses croyances religieuses. Bien avant la loi de 1905, qui a été beaucoup citée,

Nous avons accepté- je vous demande de le mettre à notre crédit -de revenir sur le terrain du droit, comme le rapporteur nous a demandé de le faire. Mais vous ne nous avez pas donné les explications que nous vous demandions. Vous ne nous avez pas expliqué les

par vous en commission mixte paritaire est devenue fondamentale et indispensable. Quelle est votre motivation profonde ? Vous nous

ont un lien ténu avec la République. Ces enfants sont scolarisés à l'école de la République, là où on forge le creuset de la société. Si nous portons l'anathème sur ces familles,

politiquement correcte interdit de tenir des débats sur la prévention de la radicalisation. Monsieur le ministre, vous avez toute ma confiance. Je sais le combat que vous menez pour la laïcité à l'école,

alors que, outre-Atlantique et dans le monde anglo-saxon en général, le lieu par excellence de la liberté individuelle, c'est la société civile. La laïcité

sens des responsabilités. Quel que soit le vote que vous ferez dans un instant, nous avons à souligner ces éléments d'unité. Il est très important en effet de dire qu'il existe un contrat social français, qui est un contrat spécifique. S'il y a un point dont on doit se réjouir, c'est qu'au fil des décennies

d'une manière qui ne soit pas apeurée mais constructive et volontariste, la supériorité de la vision républicaine du contrat social. C'est bien ce genre de choses qui se jouent là. Croyez bien que, sur ces questions, chacune de mes prises de position, aujourd'hui comme hier et comme demain, est inspirée par ce que je vois sur le terrain ; les réponses que je donne me semblent appropriées sur un plan pratique. Or, précisément, sur un plan pratique, je ne pense pas que cette proposition de loi fasse avancer ce que nous souhaitons en matière de laïcité, de lutte contre le communautarisme et de lutte contre la radicalisation. Je voudrais que nous ayons ces trois sujets à l'esprit. La lutte contre la radicalisation est par définition un sujet d'unité nationale ; elle concerne chacun des services publics, et l'éducation nationale y prend largement sa part en ce moment, même si l'on doit toujours être

évidemment les directeurs d'école dans les mesures qu'ils souhaiteront prendre pour éviter tout prosélytisme. D'une certaine façon, il vous sera démontré que nous pouvons lutter contre le prosélytisme et pour la laïcité avec les outils juridiques dont nous disposons aujourd'hui. Personne ne

Nous allons procéder au débat sous la forme d'une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents. Je rappelle que l'auteur de la demande dispose d'un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente. À l'issue du débat, le groupe auteur de la demande

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, si nous avons demandé la tenue de ce débat, c'est parce que nous estimons que le Gouvernement distille continuellement le discours de la peur. Ce faisant, il court derrière l'illusion du tout-sécuritaire et met en péril l'équilibre entre libertés publiques et sécurité. Dans ce monde dangereux, le plus grand péril est peut-être celui de la remise en cause de notre idéal de liberté, car ce monde est aussi celui où les progrès technologiques permettent un contrôle de chacun à chaque instant. Mes chers collègues, cette liberté, pour s'exprimer, s'appuie sur l'État de droit, c'est-à-dire un État qui protège les individus face à l'arbitraire en soumettant la puissance publique à de puissants contrôles, notamment la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Dans ce cadre, un État de droit a, bien sûr, besoin de forces de l'ordre, et je tiens à rendre hommage à l'action des hommes et des femmes qui ont choisi de passer, voire de risquer, leur vie pour nous protéger ; je salue leur engagement, et je me range à leurs côtés quand, à l'instar de tant d'autres agents publics, ils hurlent leur désarroi face à leurs conditions de travail indignes. Mais cela ne doit pas nous rendre aveugles au fait que nous assistons à l'institutionnalisation de la machine sécuritaire, au détricotage progressif de nos droits, au recul constant de la place du juge par rapport à celle du préfet. Oui, ce recul est constant Où en sommes-nous ? Vous avez accepté l'assignation à résidence sans intervention d'un juge. Quel bilan tirer de l'état d'urgence, qui, je le rappelle, a été instauré à un moment particulièrement grave pour notre société ? Sur les 4 600 perquisitions qui ont été menées durant la période de l'état d'urgence, seules 20 étaient liées au terrorisme et 16 seulement relevaient d'actes d'apologie du terrorisme. L'état d'urgence a occasionné l'interdiction de 155 manifestations en dix-huit mois et a servi de cadre pour ordonner 639 interdictions individuelles de manifester.

d'une particulière gravité pour l'ordre public ». C'est accepter l'idée qu'il n'est pas nécessaire de passer à l'acte pour être coupable. C'est accepter l'idée que le préfet prenne la place du juge- et nous touchons là aux fondamentaux Le Conseil constitutionnel a, fort heureusement, joué son rôle de garant et censuré ce dispositif. Avons-nous pour autant entendu ce rappel à l'ordre ? Je ne le pense pas. Vous avez accepté que la doctrine française du maintien de l'ordre devienne celle de la lutte contre les violences urbaines et que notre gouvernement considère son propre peuple comme comme son adversaire. Cela doit nous ouvrir les yeux sur les méthodes qui ont été employées depuis plus de vingt dans nos banlieues et qui, de fait, sont maintenant employées contre des manifestants de tout âge et de toutes origines sociales. Or, ces méthodes, qui nous apparaissent aujourd'hui dans toute leur violence, comment avons-nous pu accepter qu'elles soient utilisées, normalisées, légitimées, dans des quartiers de France où, désormais, l'uniforme est parfois vécu comme une menace et non plus comme une protection ? Il faut changer radicalement d'orientation et renouer les liens de notre police avec les Français. Il ne s'agit pas là de céder à l'angélisme, mais de se rendre à l'évidence : la violence engendre la violence. Nous ne pouvons cautionner les pratiques qui entretiennent les discriminations. La Cour de cassation, en novembre 2016, a relevé le caractère abusif des contrôles d'identité discriminatoires et a condamné l'État pour faute lourde. Ma collègue Michelle Meunier, élue de la Loire-Atlantique, peut témoigner de ce qui s'est déroulé sous nos yeux : comment certaines manifestations sportives ou culturelles ont servi de laboratoire de la contention, voire de la répression de la foule par les forces de l'ordre, la police finissant, à Nantes, par disperser la Fête de la musique par des des mesures disproportionnées, qui ont conduit à la chute dans la Loire de quinze personnes et à la noyade tragique de Steve. Vous avez accepté le dévoiement total de l'usage des lanceurs de balles de défense, qui blessent gravement et handicapent à vie. Depuis le début du mouvement des « gilets jaunes », vingt-cinq personnes ont perdu un oeil, cinq une main. Je voudrais ici saluer les journalistes, qui, mettant parfois en jeu leur propre intégrité physique, nous ont permis de mesurer les conséquences de cette conception du maintien de l'ordre par la répression systématique. Car qui contrôle les forces de l'ordre ? L'IGPN n'est pas indépendante, le parquet non plus, et le juge est trop peu souvent saisi. Les experts en droits de l'homme de l'ONU ont fait part de leurs inquiétudes, relevant la mise en place d'une conception nouvelle de la pratique judiciaire, celle d'une société sans vrai procès. Sont pointés du doigt le nombre élevé d'interpellations, de gardes à vue et de fouilles, l'utilisation abusive de la comparution immédiate, des audiences de nuit et des gardes à vue sans qu'aucune infraction soit constatée ou sans qu'aucune condamnation soit prononcée après coup. Malgré cela, nous offrons souvent de belles leçons de morale « à la française » à ceux qui nous alertent. Ça ... Parlons-en, justement, de ceux qui nous alertent. Vous avez accepté de sacrifier les lanceurs d'alerte, notamment les journalistes, sur l'autel complaisant du secret des affaires. Vous avez accepté de mettre en danger le secret des sources. En mai, plusieurs journalistes du et de ont été convoqués par la DGSI pour avoir diffusé des contenus relatifs à l'affaire Benalla et à l'utilisation d'armes françaises par l'Arabie saoudite au Yémen. février, faisait face à une perquisition scandaleuse ! Vous avez accepté que notre liberté d'expression soit limitée. La proposition de loi contre les contenus haineux sur internet viendra s'ajouter à la liste, alors même que nous avons observé, la semaine dernière encore, à quel point les réseaux sociaux pouvaient être des lieux de censure, après la suspension de comptes Facebook et Twitter de syndicalistes de la SNCF. Vous êtes en train de céder sur la biométrie faciale, qui va s'installer progressivement, si nous n'y prenons garde, dans notre vie quotidienne. Face à ces dérives permises par les avancées technologiques, la CNIL a de bien trop faibles moyens. Vous êtes en train de promouvoir la société de vigilance et le transfert de responsabilité de l'État vers les citoyens pris individuellement. Conséquence : ce ne sont plus les autorités qui assument, mais la société tout entière qui s'inquiète et qui, dès lors, participe à la construction des barreaux d'un espace sécuritaire toujours plus important. Toutes les digues sautent. Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble de ces dispositifs contribuent à accroître la violence dans notre société plutôt qu'à la résorber. Benjamin Franklin le disait : « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. » Mes chers collègues, un État de droit, c'est aussi un pouvoir exécutif contrôlé. Notre débat est un débat de contrôle, et nous en connaissons les limites. L'illustration en sera très certainement criante, car, quelle que soit la teneur des propos qui seront échangés ici, quelle que soit la gravité des faits exposés, qui, mis bout à bout, offrent un tableau alarmant de l'état de nos libertés publiques, le pouvoir exécutif nous répondra, certes, mais n'aura aucune obligation d'en tenir compte.

l'article XVI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose qu'une « société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » C'est sur ce fondement que nous avons construit patiemment, depuis deux siècles, notre État de droit. Cet État de droit s'est constitué autour d'institutions parlementaires et juridictionnelles. C'est le Parlement qui, tout d'abord, a su s'émanciper du pouvoir exécutif pour instituer un régime de liberté. C'est l'époque des grandes lois de la III République comme celle sur la liberté de la presse. Nous vivons encore sur ces acquis républicains, qui sont notre ADN commun. Je n'oublie pas que le Sénat fut à cette époque, notamment lors de l'affaire Dreyfus, un défenseur intransigeant de ces libertés. Je ne m'étonne pas que vous soyez encore profondément attachés à ces questions, comme en témoigne le débat d'aujourd'hui. Cet État de droit s'est aussi constitué grâce à la montée en puissance de nos juridictions judiciaire, administrative et, plus tardivement, constitutionnelle. Je ne prendrai qu'un exemple récent, avec l'introduction dans la Constitution de la question prioritaire de constitutionnalité par la révision constitutionnelle de 2008.

car je pense que, en matière d'État de droit, nous devons toujours être vigilants. Il s'agit d'une conquête permanente, et rien n'est jamais totalement acquis. Par tous les moyens, nous devons conforter et même renforcer l'État de droit. Mais faut-il considérer qu'il serait menacé en France ? en France ? En ce domaine, la vigilance n'interdit pas la rigueur et la lucidité. Oui, nous faisons face à des menaces de tous ordres, à des menaces nouvelles, à des menaces qui s'amplifient ! Le terrorisme a justement pour projet d'anéantir tout ce à quoi nous croyons ensemble

Ne nous y trompons pas. Ceux qui sèment le désordre absolu ou qui le cherchent n'ont jamais pour dessein de respecter les libertés. L'histoire en offre bien des témoignages. Face à cela, le Gouvernement est attentif à assurer le respect des libertés en trouvant des équilibres entre différentes aspirations. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'il s'agit de rendre possible le droit de manifester dans des conditions sereines en empêchant les casseurs- car c'est bien de ce cela dont il s'agit -de porter atteinte aux personnes et aux biens. Tel est aussi le cas lorsqu'il s'agit de lutter contre la propagation de la haine en ligne dans un espace numérique où le meilleur et le pire souvent se côtoient. Nous devons trouver des équilibres entre le maintien de la liberté de cet espace, mais aussi le respect des personnes en mettant fin à ce qui s'apparente parfois à des torrents de haine déversés en toute impunité.

Quant à la justice, elle demeure le fondement même de l'État de droit. Le Gouvernement s'est engagé dans une réforme de fonctionnement avec la loi de programmation de la justice afin de donner plus de moyens à cette dernière et de lui permettre d'être plus accessible à nos concitoyens. C'est également préserver l'indépendance de la justice. La loi organique de 2013 a interdit les instructions individuelles faites aux parquets. Le Gouvernement respecte scrupuleusement cet interdit. Quant aux nominations des membres du parquet, le Gouvernement propose que le Conseil supérieur de la magistrature donne désormais un avis conforme. Madame Madame la sénatrice, vous avez pris des positions très critiques faisant état d'une présidence autoritaire ou de lois liberticides. Votre droit de porter ces critiques est fondamental, et je suis heureux que vous puissiez l'exercer pleinement. C'est ce qui nous vaut ce débat aujourd'hui. Mais je crois que ce sujet est suffisamment important pour ne pas porter de jugements excessifs ou à l'emporte-pièce, car l'État de droit est une chose précieuse et fragile. Par son article V, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen affirme : « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Des lois sont votées. Certaines d'entre elles défendent les actions nuisibles à une société fragile et en proie au doute. Le Conseil constitutionnel veille à ce que les lois respectent l'État de droit. Telle est la situation dans notre pays. Je crois que nous devons en apprécier toute la réalité, car, dans bien d'autres pays, y compris parfois en Europe, tel n'est pas tout à fait le cas. Nous allons Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, suivie d'une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

En effet, l'État de droit suppose le respect de la hiérarchie des normes, l'égalité devant le droit et l'indépendance de la justice. La loi votée par le législateur peut être déclarée inconstitutionnelle par une cour qui s'appuie sur un certain nombre de principes. La réforme du 23 juillet 2008 de notre Constitution permet, sous certaines conditions, d'invoquer l'inconstitutionnalité d'une loi. C'est la question prioritaire de constitutionnalité. On peut également considérer l'État de droit d'une façon bien plus large que le seul respect de la hiérarchie des normes, en intégrant dans sa définition un contenu dont le coeur est, en France, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Constitution de 1958. Dès lors, il apparaît que la question des mesures à prendre d'urgence pour lutter, par exemple, contre les violences terroristes, met en cause ces différentes conceptions de l'État de droit. Or, dans les pays démocratiques, il est essentiel que les ennemis de la démocratie soient combattus par des moyens démocratiques. C'est même la difficulté centrale L'État de droit existe lorsque la loi votée par le Parlement est appliquée et que les décisions administratives sont rapidement exécutées. L'État de droit existe lorsque les citoyens ont confiance dans les institutions de la République et que celle-ci sait, d'une part, se faire respecter et, d'autre part, faire respecter les droits fondamentaux Pour ma part, mes chers collègues, sur ces deux points et pour ne citer qu'eux, il me semble que le doute est permis et que le recul est flagrant. Aussi prenons garde, monsieur le ministre, à cette situation, car, lorsque l'État de droit est bafoué, ce sont la cohérence et la solidarité de la nation qui sont menacées. Qu'entendez-vous faire pour améliorer cette situation

on le sait depuis deux siècles, et c'est finalement l'un des héritages des Lumières et de la Révolution française -, mais aussi et surtout de la doctrine constitutionnelle du début du XXsiècle, en particulier celle de Hans Kelsen. Dans notre pays, nous avons désormais un édifice juridique très robuste. L'institution du Conseil constitutionnel en 1958, sa décision de 1971 sur la liberté d'association, sa saisine ouverte à soixante parlementaires- réforme que l'on doit au Président Giscard d'Estaing -et, enfin, l'introduction de la QPC en 2008 tout cela a contribué à ce que notre bloc de constitutionnalité soit protégé et respecté. La loi doit respecter la Constitution, vous le savez mieux que moi encore. Elle doit aussi respecter les conventions internationales, singulièrement la convention européenne des droits de l'homme. Il appartient ici à toutes les juridictions d'assurer ce respect, ce que les juges judiciaires depuis 1975 et les juges administratifs depuis 1989 font. C'est aussi l'une des conditions absolues de notre État de droit. Il s'agit même d'une certaine façon de sa clé de voûte. Le Gouvernement est toujours attentif à ces données juridiques, comme le Parlement d'ailleurs. Il ne le serait pas que les juridictions, en particulier le Conseil constitutionnel, nous rappelleraient à l'ordre, comme elles le font parfois à bon escient. La parole

Notre Constitution prévoit que le juge judiciaire est garant de nos libertés individuelles. L'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme garantit, quant à lui, le droit à un procès équitable, dont le principe du contradictoire est un des fondements. Or nous assistons actuellement à un inquiétant glissement des prérogatives du juge judiciaire vers l'exécutif et l'administration, mais aussi à plusieurs atteintes aux droits de la défense, qui sont particulièrement inadmissibles et inquiétantes pour nos libertés. À ce titre, j'évoquerai les pratiques relatives à des personnes étrangères « entendues » en visioconférences effectuées depuis un commissariat dans le cadre d'un appel de la décision du juge des libertés et de la détention prolongeant leur enfermement, l'attente d'une procédure d'éloignement. Cela s'est produit dans un commissariat, un établissement de police, dépendant du ministère de l'intérieur, qui jouxte le CRA d'Hendaye au Pays basque ! Plusieurs associations et syndicats d'avocats ont dénoncé ces audiences scandaleuses « conçues dans le seul but de faire l'économie des escortes policières et « tenues en violation des principes les plus essentiels régissant les débats judiciaires dans un État de droit ». Si les vidéoaudiences, sans consentement des intéressés, ont été malheureusement introduites avec le vote de la loi Collomb relative à l'asile et à l'immigration, il n'en demeure pas moins que l'article L. 552-12 du prévoit à cette fin des « salles d'audience ouvertes au public » et la « confidentialité de la transmission ». Or, en l'espèce, un commissariat n'est pas une salle d'audience remplissant ces conditions ! Ces vidéoaudiences semblent donc dépourvues d'une base légale. Comment rendre une justice impartiale depuis des locaux de police et en dehors d'un bâtiment du ministère de la justice ? Comment rendre la justice sans respecter les conditions de son exercice, de son impartialité et le droit de la défense ? Monsieur le ministre, dans un climat où le justiciable manifeste de plus en plus de méfiance à l'égard du système judiciaire, comment peut-on justifier de telles dérives ?

Le code de procédure pénale décrit précisément les cas dans lesquels des personnes peuvent être placées en garde à vue. Il s'agit, principalement, de conduire l'enquête et d'empêcher que l'infraction ne se poursuive. C'est une mesure essentielle au travail d'investigation, qui a son équivalent dans tous les systèmes juridiques. vue est soumise enfin au contrôle des juridictions de jugement lorsque la procédure est présentée au tribunal. Vous posez la question du recul en France de l'État de droit en raison d'un recul du juge dans ce domaine. Je puis vous garantir qu'il n'en est rien. L'emploi des moyens coercitifs est très encadré et le contrôle du juge est omniprésent, que ce juge soit le juge national ou parfois le juge européen.

consubstantielles à notre démocratie. Ce rappel est salutaire : notre État de droit n'est pas un acquis qu'il nous suffit de revendiquer par réflexe, sans conscience ni vigilance. Il doit être protégé en permanence et affermi contre tous ceux qui abusent de ses valeurs pour prêcher l'intolérance et tenter de miner nos libertés. Oui, notre République est le fruit d'une histoire complexe, d'oppositions, de luttes, comme de moments d'unité nationale lorsque l'essentiel est en jeu ! La démocratie représentative en est l'incarnation, certes imparfaite, mais sûrement la plus poussée pour que s'expriment les composantes du corps social. Le Parlement vote la loi, dans les conditions fixées par la Constitution de 1958, mais encore faut-il qu'il dispose de toute l'information utile pour délibérer en connaissance de cause. Or notre société tend vers toujours plus de complexité et d'informations à trier et à analyser. J'ajoute que la Constitution favorise structurellement la concentration par le pouvoir exécutif de la masse critique de données nécessaires pour légiférer. Je pense, par exemple, aux données de fiscalité locale, qui seraient indispensables au représentant des collectivités territoriales qu'est le Sénat. C'est enfin peu dire également que les études d'impact sont des coquilles vides en ce qu'elles n'engagent pas à grand-chose, puisque seul leur formalisme fait grief. Ma question est donc simple : comptez-vous améliorer l'information préalable du Parlement, en lui donnant réellement accès à davantage de données, afin de nourrir ses travaux et d'éclairer ses votes ? monsieur le ministre parlementaires en amont des débats législatifs. Il me semble qu'on essaye de progresser, puisqu'un agenda prévisionnel sur trois mois est envoyé au Sénat pour faciliter le travail en amont et que nous avons pu, dans certains cas- c'est au président du groupe du RDSE que à la construction avec les sénateurs. Je pense, par exemple, à la conférence de consensus qui s'est tenue sur le logement, initiative proposée par le Sénat pour préparer le projet de loi sur le logement. Deuxièmement, vous m'interrogez sur les études d'impact et leur caractère parfois imparfait, incomplet

de la réforme envisagée. Ce sont des objectifs mesurables, tournés vers les Français, pour partie qualitatifs et aisément compréhensibles par tous : faciliter l'information des sénateurs et améliorer le suivi

indéniablement, l'État de droit est mis à mal au sein de la nation. Qu'est-ce qu'un État de droit ? Un système institutionnel dans lequel la séparation des pouvoirs est de mise.

avec le mouvement social des « gilets jaunes », à l'encontre des lycéens de Mantes-la-Jolie ou quand le jeune Steve a disparu. Depuis plusieurs années, tant les exécutifs successifs que la majorité conservatrice du Sénat utilisent la loi pour porter atteinte à de nombreux droits fondamentaux. En 2017, un projet de loi a fait entrer dans le droit commun des dispositions de l'état d'urgence. En avril et en octobre 2019, des propositions de loi sont venues gravement porter atteinte aux droits à manifester et à s'exprimer dans l'espace public. Peu à peu, nous entrons dans une société de la répression permanente. Les droits inhérents à une démocratie moderne sont mis à genou au nom de la lutte contre le terrorisme et du maintien de l'ordre public. Alors que tout semble désormais permis en matière sécuritaire, ma question est simple, monsieur le ministre : quand les pratiques de nos forces de police seront-elles encadrées, sur le modèle de la « désescalade » dans les manifestations appliquée en Allemagne et dans les pays scandinaves ? monsieur le ministre assez régulier à la violence dans les manifestations, c'est un problème pour l'État de droit. La menace qui pèse sur les journalistes dans leur travail, c'est une menace contre l'État de droit. Les violences à l'endroit des policiers ou des forces de secours, c'est une menace contre l'État de droit.

se dote de moyens et d'outils pour rétablir l'État de droit et protéger nos citoyens, y compris dans leur droit de manifester. Je vous rappelle que nous sommes profondément attachés- cela a été rappelé à plusieurs reprises -à la liberté de manifestation. Ce droit s'inscrit dans les racines de notre démocratie, c'est d'ailleurs un droit et une liberté fondamentale.

inouïe ont été commis à Paris ou en région. Chacun a pu le mesurer : cela n'a plus rien à voir avec le fait d'exprimer son opinion sur la voie publique. Les parquets ont exercé leurs prérogatives, conformément à la loi. Des manifestants qui commettent des actes délictuels- pillages, violences -contre les forces de l'ordre ne sont plus des manifestants et doivent être poursuivis conformément à la loi. Garantir l'État de droit, c'est garantir la possibilité de manifester publiquement. Je ne voudrais pas que, par notre incapacité à empêcher les Black Blocs d'agir, nous privions les manifestants pacifistes du droit à manifester. C'est bien dans ce cadre-là

la sécurité doit nous permettre d'exercer nos libertés et non de les restreindre. Vous avez parlé des « gilets jaunes » et de leur violence. Je crois que vous les confondez avec les Black Blocs

mais, curieusement, les Black Blocs n'ont pas souvent été arrêtés ... Notre population est meurtrie par plusieurs mois de contestation sociale. Le rôle de l'État de droit est de permettre à nos concitoyens d'exercer leur liberté d'expression et de manifester. Les manifester. Les entraves se multiplient ces derniers mois. Je crains, hélas ! que nos institutions ne puissent bientôt plus garantir liberté et sérénité aux mouvements sociaux populaires

Afin de parer les menaces, des mesures ont été prises. Le gouvernement précédent y a largement contribué, notamment avec l'importante loi relative au renseignement de 2015 et un état d'urgence prolongé. La majorité actuelle poursuit cette démarche, et certains sont inquiets de voir la liberté de plus en plus contrainte au profit de la sécurité. Il est vrai que nous voyons dans le domaine de la sécurité, comme dans les autres, proliférer une inflation législative toujours plus difficile à maîtriser. « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », disait Montesquieu. La profusion permanente de nouvelles règles fait peser un risque sur l'État de droit. Nul n'est censé ignorer la loi, mais qui peut prendre connaissance et retenir la soixantaine de lois promulguées chaque année ? le groupe Les Indépendants est convaincu que nous devons collectivement veiller à limiter la production de nouvelles normes et à ce que les lois restent de portée générale et visent à s'appliquer à tous. à tous. Cela nous permettrait d'améliorer sensiblement la stabilité du cadre juridique de nos concitoyens, mais aussi la connaissance des libertés et des devoirs de chacun. À l'heure actuelle, certaines normes créent de nouveaux dispositifs censés être plus adaptés aux situations nouvelles. Mais nous constatons bien souvent qu'un dispositif préexistant, de portée plus générale, pourrait suffire à régler les difficultés récentes s'il était effectivement mis en oeuvre.

Aucun esprit, aussi puissant soit-il, même s'il avait les capacités d'un Pic de la Mirandole, n'est en mesure aujourd'hui de maîtriser tout notre corpus législatif. Vous le soulignez à juste titre : lutter contre l'inflation législative est au fond un vieux combat. Chacun s'y est attaqué à sa façon, quelles que soient les majorités. Le Sénat a pris des initiatives heureuses, par exemple, en déclarant irrecevables de manière systématique les amendements non normatifs, les cavaliers divers ou réglementaires. Mais cela ne peut suffire, et le chantier est immense, car nous partons de loin. Des solutions plus fortes pourraient être trouvées, je suis d'accord avec vous. Si la Constitution de 1958 établit une distinction plus stricte entre la loi et le règlement, c'est aussi pour préserver le caractère simple, lisible et surtout général de la loi. Nous devons retrouver collectivement cet esprit et cette inspiration initiale. Il faut être conscient que voter des lois plus générales, c'est aussi donner plus de latitude aux juges pour régler au quotidien les litiges. Cela a toujours été l'office

Ainsi s'exprimait Chateaubriand, lui qui avait tout connu des horreurs de la terreur révolutionnaire, de l'autoritarisme impérial et de la réaction de Charles X. Il nous rappelait que sans liberté les citoyens ne sont plus que des individus isolés, isolés, face à un État porté par nature à réduire la liberté au nom de l'efficacité. Certes, la France de 2019 n'est plus celle de 1848. La France est évidemment un État de droit, donnant vie à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'elle est si fière d'avoir rédigée. Néanmoins, depuis quelques décennies, notre législation tend davantage à multiplier les interdits, à accroître la répression et à banaliser les exceptions plutôt qu'à proclamer et à protéger de nouvelles libertés. Nous réduisons largement les libertés des individus dans la société en contrepartie d'une sécurité qui n'est pas toujours bien vécue. Que la violence et la haine soient blâmables ne fait aucun doute. Que le terrorisme soit le fléau de l'époque pour lequel aucune pitié n'est permise, assurément. Mais cela ne doit pas se faire au mépris de nos libertés que détestent tant ceux que nous combattons. Force est néanmoins de constater que le recul des libertés se fait par petites touches. Pour ne citer que deux exemples, est-il pertinent de demander au juge de définir dans l'urgence ce qu'est une « fausse information » et ce qui ne l'est pas ? Est-il opportun de réinstaurer une sorte de délit d'opinion comme le préconise la relative à la répression des discours de haine sur internet ? Cette proposition de loi fera des gestionnaires de réseaux sociaux des censeurs arbitraires, sans légitimité démocratique. La liberté a un prix : celui d'être blessé, révolté et atteint par les opinions contraires.

en arriver à instaurer des mécanismes qui restreindraient les libertés d'expression, mais il importe aussi de sanctionner ce qui relève d'un délit. On ne doit pas impunément pouvoir appeler dans l'espace virtuel à la haine raciste, à l'antisémitisme, à l'homophobie ni proférer

Guy Carcassonne l'affirmait : « L'emploi de la force publique ne peut se faire que dans le respect du droit, et c'est le fait que l'État se plie à cette exigence qui définit justement ce qu'on appelle l'État de droit Cette idée figure à l'article XII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. l'État de droit comme rempart à l'arbitraire, à l'État de police qui ne connaît pas d'autre limite à sa volonté ou à son action que celle de ses forces. Après l'attaque de la préfecture de police, le Président de la République a affirmé que les institutions seules ne suffiront pas à venir à bout de l'islamisme souterrain. Il a appelé « à bâtir une société de la vigilance exigeant de chaque citoyen qu'il apporte son concours à la force publique. Ces déclarations ont probablement justifié le présent débat. Si elles interrogent, elles sont surtout révélatrices d'une impuissance de l'État à faire respecter le droit, à faire cesser les atteintes et les provocations contre la République. Cette crise de l'État de droit ressort, tout d'abord, de son incapacité à garantir la sécurité sans entraver la liberté. La sécurité n'est pas une liberté, mais c'est l'une des conditions de l'exercice de nos libertés. Pendant la crise des « gilets jaunes », la réponse de l'État a été de dire : n'allez pas manifester, car vous ne serez plus en sécurité. Comment en est-on arrivé là ? Un an et demi après l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les ex-zadistes sont toujours présents et les tensions demeurent. Cette crise existe aussi au plus haut de l'État, lorsque l'exécutif critique une mission d'information qui témoigne pourtant de l'indépendance d'une assemblée parlementaire dans l'exercice de son devoir de contrôle, ou encore lorsque la présence d'un juge d'instruction pourrait dépendre des résultats électoraux. Je conclurais par une citation du général de Gaulle Plus le trouble est grand, plus il faut gouverner ! » Monsieur le ministre, quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour que l'État de droit ne recule plus en France ? La parole est

peut recourir dans certains cas- et dans certains cas seulement -à la force. L'État de droit doit être protégé contre tous les actes qui entendent y porter atteinte. Je suis d'accord avec vous : pour que l'État de droit existe, il est nécessaire que l'État dispose des moyens juridiques, matériels et humains lui permettant de l'exercer. C'est d'ailleurs de ces moyens dont nous

revanche, je suis moins d'accord avec vous quand vous parlez de la séparation des pouvoirs. Lorsqu'un ministre de la justice appelle à respecter la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice au moment de la création d'une commission d'enquête, il s'agit tout simplement de la stricte application de l'ordonnance du 17 novembre 1958.

En 2015, compte tenu d'une situation dramatique, nous avons dû nous résoudre à déclarer l'état d'urgence et à donner à l'administration des compétences auparavant dévolues au seul juge du siège. auquel vous appartenez, monsieur le ministre, a décidé que ces mesures exceptionnelles devaient entrer dans le droit commun, confortant ainsi, en particulier, le rôle du parquet, du procureur, en cas de mesures administratives prises à titre préventif. En 2018, la conjugaison de votre doctrine et de l'évolution de la doctrine du maintien de l'ordre face à la crise des « gilets jaunes », marquée par votre volonté d'appliquer aux manifestants des dispositions inspirées de la lutte antiterroriste en donnant aux préfets des pouvoirs de prévention et d'interdiction de manifester vis-à-vis de personnes non condamnées par un juge,

monsieur le ministre,

le maintien de l'ordre et l'usage juste et proportionné de la force publique sont seuls légitimes dans une démocratie, afin de de rétablir la paix publique lorsque des troubles sont causés et à l'égard de ceux qui ne respectent pas le cadre légal de la manifestation publique. La doctrine de maintien de l'ordre établie par le Gouvernement s'inscrit

les élus ayant participé à cette consultation, 92 % affirment avoir été victimes d'incivilités, d'injures, de menaces ou d'agressions civiques. Or ils ne sont que 37 % à avoir saisi la justice, et 21 % seulement des plaintes ont abouti à la condamnation pénale des fautifs.

Si l'État de droit s'impose à l'État pour la protection des libertés individuelles et des droits de l'homme, il s'impose également aux individus, qui ne peuvent en faire un totem. Car l'État de droit n'est pas une orientation politique ou idéologique, mais consiste en l'application des règles de droit.

fait, la défiance généralisée, synonyme de manichéisme croissant, ne saurait justifier qu'on se soustraie aux règles de droit pour répondre aux fractures sociales et territoriales qu'elle dénonce. Ce serait apporter de mauvaises réponses à de bonnes questions et affaiblir encore plus le fonctionnement apaisé de notre démocratie.

ou leur permanence. Ainsi, la garde des sceaux prépare une circulaire, qui sera diffusée dans les prochains jours à l'ensemble des procureurs généraux et des procureurs de la République, afin de rappeler que les infractions commises contre les élus, qu'ils soient dépositaires de l'autorité publique, comme les maires, ou chargés d'une mission de service public, comme les parlementaires, sont aggravées du fait de leur qualité ; que la réponse pénale, si elle doit être adaptée aux faits et à la personnalité des auteurs, doit être systématique, systématique, après défèrement des mis en cause dans les cas les plus graves ; et que les élus victimes doivent être systématiquement tenus informés des suites données à leur plainte. Plus largement, le dialogue entre les élus, les forces de police et les parquets, déjà permanent, doit être une priorité, car, au-delà du meilleur traitement de la délinquance qu'il permet, il doit aider à comprendre les préoccupations et les alertes et, ainsi, à mieux prévenir les atteintes aux élus,

c'est l'abandon de l'État de droit en zone rurale sur des milliers d'hectares, la démission des pouvoirs publics face à la violence de groupuscules, des voies publiques confisquées au détriment de la circulation : bref, une zone où la République s'est effacée pendant plusieurs années. En 2016, les manifestations violentes à Nantes ne furent ni interdites ni autorisées

le même Édouard Philippe qui, le 17 janvier 2018, annonça l'abandon définitif du projet, faisant fi de plus de 170 décisions de justice favorables. Sous

nommait commissaire enquêteur un propriétaire foncier pour ouvrir les droits à construire : aucun maire ne pourrait l'admettre, ni l'État d'ailleurs avec son contrôle de légalité. Pour couronner le tout, un représentant de l'État, préfet de région, est allé trinquer avec les zadistes à l'annonce de l'abandon du projet ... Chaque fois que le politique manque de courage, c'est l'État qui s'affaiblit. Et l'État qui faiblit, c'est le recul du droit ! Très bien

de l'aéroport actuel en direction de l'une des plus grandes zones humides de France et le sacrifice d'habitants de la banlieue nantaise, notamment ceux de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu, qui subiront

et même les médias traditionnels. D'ailleurs, ceux qui souhaitent nuire à la démocratie commencent souvent par s'en prendre à la presse. Voici ce que disait un de nos illustres prédécesseurs, Victor Hugo : « La liberté de la presse à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une c'est attenter à l'autre. » Le dernier rapport de Reporters sans frontières fait état, pour la seule année 2018, de la mort de 80 journalistes, dont 49 assassinés en raison de leur profession. En dix ans, ce sont 702 journalistes qui ont trouvé la mort dans ces conditions. Par ailleurs, 348 journalistes sont en détention et 60 gardés en otage. Voilà l'état de la presse dans le monde

la situation économique de la presse se dégrade, laissant apparaître des concentrations inédites, avec des risques pour l'indépendance des titres, et des achats d'éditeur sans respect des rédactions, malgré nos lois. De plus en plus de journaux et de chaînes peinent à produire de l'information par manque de moyens. Actuellement, nous nous débattons face aux Gafam pour que la presse bénéficie de la valeur qu'elle crée. aussi d'ordre international, avec la divulgation par certains États ou personnes affiliées d'infox qui influencent l'issue d'élections ou de référendums et, plus généralement, s'attaquent au débat démocratique. Elles sont, enfin, d'ordre sociétal, car une parole violente s'exerce contre les journalistes, ouvrant la voie à des attaques physiques contre ceux qui se rendent sur le terrain.

monsieur le ministre,

au regard de la loi, l'équité dans l'application de celle-ci, la séparation des pouvoirs, la participation à la prise de décision, la sécurité juridique, le refus de l'arbitraire et la transparence des procédures. En d'autres termes, peut se prévaloir de ce nom un État dans lequel le droit s'impose à tous. Or de nombreuses situations nous portent à croire que notre État de droit s'est étiolé et que certains mouvements minoritaires, souvent radicaux, pèsent davantage dans notre démocratie que la majorité silencieuse.

Le 9 octobre dernier, l'instance de coconstruction, selon les termes devenus habituels, chargée de trouver une alternative à la retenue d'eau de Sivens a décidé de lancer un complément d'étude sur les besoins en eau dans la vallée du Tescou. Si l'on peut se

qui ne veulent pas forcément du bien à la République ni à la loi, donnent des mots d'ordre de désobéissance civile consistant, en vérité, à empêcher les autres d'exercer leurs libertés. actions sont souvent pacifiques ; mais, parfois, quelques individus, peut-être intellectuellement mieux armés, incitent les uns ou les autres à un peu plus de violence ou sont le ferment

Cette critique de la démocratie représentative conduit trop souvent à ignorer la loi, voire à la combattre, au nom d'une conscience individuelle qui surplomberait la délibération démocratique.

pouvons-nous considérer que, face à l'un des principaux défis de notre temps, le terrorisme, notre démocratie peut rester forte sans se renier elle-même ? Sur ces travées, visiblement, la réponse va au-delà de la gauche. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous remettre un livre, un livre, écrit par un de vos camarades de combat- puisqu'il a écrit les statuts du parti En Marche. L'auteur conteste cet accommodement cet accommodement avec le « surveiller plus » et le « châtier davantage », après le terme de la peine s'il le faut, pourquoi pas avant même que le crime ne soit commis et en se passant parfois des droits de la défense. La surveillance peut s'étendre graduellement,

! Seulement, nous avons un ministre de l'intérieur qui ne pense pas la même chose. Selon lui, « rien ne menace la liberté si ça permet de lutter efficacement contre le terrorisme ». Or l'expérience prouve qu'un régime ne peut rester démocratique que si la liberté est soigneusement garantie, y compris en limitant l'État. Vous en avez eu de nombreuses illustrations

mettre des semaines à rendre compte des conditions de la mort de Steve, l'homme tombé dans la Loire le soir de la Fête de la musique, de ne toujours pas nous donner les conclusions de l'IGPN sur les très nombreuses violences policières qui ont été constatées au moment des manifestations des « gilets jaunes

-toute tentative de contrôle, qu'il s'agisse du contrôle parlementaire- le président Requier l'a évoqué -, comme au moment de la commission d'enquête dite Benalla, ou du contrôle citoyen, au travers de la proposition de loi référendaire sur la privatisation d'ADP, dont on ne peut pas dire que l'État

face à la montée des extrémismes politiques dans notre pays. Ce que nous cédons, ce que vous cédez aujourd'hui par facilité, ou parfois peut-être par ignorance, c'est l'esprit même de nos institutions